La séance s'est reprise les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunis à 19 heures sont consultables sur le site du Sénat. Elles sont considérées comme adoptées en l'absence d'observation, d'ici la fin de la séance de ce soir. J'informe le Sénat que les candidatures ont été publiés pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du règlement sur les directives de négociations en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, d'une part et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, présenté par Monsieur messieurs Pascal Alizart et Didier Marie demande de la commission des affaires économiques de la commission des affaires européennes et la commission des Affaires étrangères. Bien, mais Monsieur le ministre. Mesdames, monsieur le président, Mesdames, messieurs les rapporteurs donc dans la discussion générale, la parole est à monsieur Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, en remplacement de messieurs Pascal Alizart et de monsieur Didier Marie, auteur de la proposition de résolution et rapporteur pour avis de la commission des affaires européennes.

c'est la première fois qu'en séance publique, nous sommes amenés à débattre de mandat de négociations concernant des accords de libre-échange avant avant leur adoption par le Conseil notre assemblée est ainsi en mesure de faire. Vouloir en amont des négociations les points essentiels sur lesquels souhaite être entendu par la commission par le Conseil, mais aussi Monsieur le Ministre, par le gouvernement, notre démarche. Prend une signification particulière à l'heure où les futurs accords de libre-échange pourrait ne plus être systématiquement soumis à la fin des négociations au ratification des parlements nationaux. C'est là toute la conséquence de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, en mai dernier, comme Singapour qui à déterminer ce qui, dans ses accords relève de la compétence exclusive de la Commission ou des compétences partagées avec les États membres, d'où l'importance pour les parlements nationaux, d'être impliqué ou de s'impliquer, de même, comme c'est le cas ce soir le plus en amont possible des négociations, d'où aussi l'importance pour nous d'être également associés de façon régulière et transparente au déroulement des négociations qui s'ensuivront faudrait rappeler que dans la commission d'accord tant que la commission Affaires économiques ont toujours été extrêmement attentive aux demandes des différents collègues qui, au travers des propositions de résolution souhaitée, je dirais que ces débats

rapporteur pour avis, donc je vous prie d'excuser l'absence, aujourd'hui ils sont retenus à Vienne pour je dirais le au niveau de l'organisation de de de l'OSCE, le rapport de notre collègue Anne-Marie Bertrand, au nom de la commission des affaires économiques, a fort bien approfondi les enjeux, de quoi s'agit-il ces projets d'accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande concerne 2 pays qui pourrait être géographiquement très éloignés, nous sont proches sur le plan des valeurs démocratiques comme de la conception multilatéralistes des relations entre État, nous entretenons déjà avec des partenariats politiques et des Liens commerciaux significatifs, la proposition de résolution européenne, affirme un certain nombre de principes et de garde-fous, ils doivent bien sûr valoir pour ces 2 accords mais aussi guider les négociations sur toute autre accord de même nature et la politique commerciale européenne en général, j'en vois 4 la transparence, l'équilibre, la réciprocité et l'exigence normative d'abord la transparence sur ce point, nous revenons de loin, vous le nous devons avoir l'on était de reconnaître que de réels progrès ont été accomplis, ils sont venus de la Commission européenne elle-même récemment encore de notre président, Jean-Claude Juncker, ils sont aussi venus du gouvernement qui a su associer parlementaire et société civile aux avancées ou au blocage des négociations de certains accords passés, on doit aussi s'progrès au mouvement d'opinion qui ont pu prospérer sur l'opacité qui était jusqu'alors la règle, ils ont mis à jour des craintes souvent légitimes, parfois aussi exagérée que suscitait cette pratique du secret, ça vient aussi, je l'ai dit à l'instant du Sénat en particulier qui travers de son souhait de prospective et de son n'attachement au territoire a bien compris l'intérêt si vous voulez de l'équilibre, ensuite il s'agit de faire preuve d'une vigilance constante, en particulier sur les produits agricoles sensibles au 1er rang desquels, en l'espèce les viandes bovines et ovines, mais aussi les sucres spéciaux. La promotion de résolution européenne s'appuie sur ce que le Sénat depuis longtemps mis en avant, à savoir que l'accord après accord, les mêmes menaces s'accumulent sur les mêmes filières déjà fragilisés dans nos territoires, nous avons d'ailleurs à l'esprit en toile de fond les ultimes marbré Trajan courent sur le corps sur Marco sourd cela n'exonère certes pas certaines de ces filières, de procéder à d'opportunes Restructuration, je n'ai jamais eu, je dirais, j'ai toujours eu plus exactement, l'occasion de le rappeler, notamment la filière bovine au travers des différents acteurs, ce n'est pas leur faire injure, ni les provoquer, parce que nous sommes, avec à leur côtés en la matière, tant en ce qui concerne la redéfinition et le redimensionnement du fonds d'adaptation à la mondialisation, que de la structuration proprement dite de la filière remontera vers de la création des Opel production carrément par bassin il y a beaucoup d'autres critères, il reste que l'on se trouve là, au coeur de l'ambiguïté de la mondialisation, ses bénéfices sont globaux, mais ces effets négatifs sont locaux, ils nous régions nos campagne des exploitations des hommes et des femmes, c'est aussi pourquoi nous voulons que les crédits de la politique agricole commune soit préservés dans le prochain cadre financier pluriannuel les uns et les autres, nous nous sommes exprimés en la matière et et j'avoue que nous arrivons à une période un peu cruciale : j'aimerais bien que la France soit aussi le déterminer que le fut par le passé en la matière. L'Union européenne a créé un fonds d'ajustement à la mondialisation, c'est en effet de cela qu'il s'agit, permettent aux filières transition de s'ajuster aux enjeux d'un commerce ouvert malheureusement ce fonds n'est ni dotés ni structurée à la mesure de cette ambition, la résolution propose d'aborder ce. Sujet de fond, regardez comment il fonctionne pratiquement à hauteur de 150 millions d'euros et ne concerne que les entreprises. Qui se voit je dirais fragilisé par ces accords avec un nombre important de licenciements mais jamais, en aucune façon on aborde, au travers de ces fonds d'justement de la mondialisation, la problématique purement agricole la gestion attentive et prudente des contingents aux partenaires le déclenchement rapide de mesures de sauvegarde efficace la en la matière, il faut reconnaître que, entre l'Union européenne et les États-Unis. Même si cet accord ne concerne pas les États-Unis, pays fédéral par essence, les États-Unis, la fameuse mesure de mémoire 623 qui en quelques minutes, permet au travers de la clause de sauvegarde, de fermer les frontières, je dirais américaine en Europe, il faut l'accord des 27 États-membres pour mettre en place ces clauses de sauvegarde et ça demande souvent. Quel que moi et comme nous sommes, si vous voulez, encore une fois, à 27 tout le monde n'est pas toujours d'accord sur ce sur La réciprocité 3ème Focus, il y a sur ce point, beaucoup de terrain reconquérir en particulier sur l'accès aux marchés publics de pays partenaires, l'Union européenne a longtemps été très généreuse trop généreuse, voire quelquefois naïve, au contraire, de bien des pays avec lequel nous saluons ou Celeron des accords de libre- échange, et là encore, je voudrais vous rappeler, Monsieur le Ministre, que tant la commission des affaires économiques que la Commission de faire européennes on a contribué à la réflexion en la matière pour muscler la politique européenne sur ce point et faire en sorte que l'Europe, encore une fois, ne soit pas au moins naïve l'exigence normative, enfin, la proposition de rappel, le niveau d'exigence européen matière sanitaire et phytosanitaire pour les produits agricoles et agroalimentaires doit rester le même s'ils le font, il doit même être améliorés, mis à jour régulièrement, sans que les accords de libre-échange n'y fasse obstacle de même en est-il des normes sociales et environnementales, la résolution à cet effet, demande que les dispositions sur le développement durable soit opposable et contraignante dans le cas de procédures de règlement inter-étatiques adapté en conséquence le nécessaire maintien de ce droit des États Alisher légiférer amène aborder la question de la protection des investissements, les 2 propositions directives de négociation ne prévoit pas de dispositions spécifiques de règlement des différends entre investisseurs et États l'absence d'une telle mention qui aurait conféré un caractère mixte aux 2 accords ça se cri comme j'ai déjà mentionnée dans la logique de la vie, la Cour de justice, la Commission en a tiré les conséquences en privilégiant une procédure de négociation et de conclusions accélérer accélérer in fine et celle-ci n'appliquera, outre la Commission elle-même que le Parlement européen et le Conseil, celui-ci se prononçant à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité, c'est la raison pour laquelle, moi j'estime que. Les débats très en amont sont précisément nécessaire, tout simplement pour définir un cahier des charges à l'adresse du négociateur et du seul négoce. Auteur en l'occurrence Madame Maelström, le négociateur de je dirais de du de la Commission nous sommes pourtant essentiel qu'en cas de litige les partis investisseurs européens Néozélandais, Australiens puissent, si elles le souhaitent se tourner vers un système juridictionnel spécifique, même si les systèmes judiciaires nationaux Néozélandais et Australiens obéissent à des règles, des standards comparable au surplus la configuration nouvelle du système juridictionnel des investissements a opportunément améliorer et moraliser l'ancien système d'arbitrage privé nous souhaitons donc parallèlement à la négociation de 2 accords de libre-échange, la Commission engage des accords particuliers pour la protection des investissements. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a, je crois, dans cette assemblée une majorité favorable à une politique commerciale européenne ambitieuse pour peu, pour peu qu'elle respecte les principes d'équilibre et de réciprocité, nos entreprises peuvent y valoriser leur intérêt offensif qui sont nombreux, y compris parfois dans certains secteurs agricoles. En tant qu'élu de Normandie, je n'ose pas vous rappeler que l'accord sur le CETA aura permis d'abaisser les barrières tarifaires sur un certain nombre de fromages de près de 140 aura permis une reconnaissance, si vous voulez de près de 43 ou 45 indication géographique de provenance, mais ceci n'exclut pas, entre guillemets, une grande vigilance sur ce type je dirais d'accord pour la bonne et unique raison c'est que tous les toutes les filières et tous les agriculteurs ne sont pas armés, si vous voulez pour affronter, je dirais, les grands marchés internationaux, c'est là encore une fois, je me répète, l'intérêt du fonds d'adaptation à la mondialisation et l'intérêt aussi je, je, je dois l'avouer Monsieur le Ministre le de la République n'avaient-ils pas émis l'idée d'accorder pratiquement ou de ou d'ouvrir une ligne budgétaire de 5 milliards d'euros à l'adresse des filières qui voulait se réformer et se moderniser, hé bien il y a là si vous voulez un débat qu'il faudra qu'un que que l'on ouvre sur ce point parce que, là encore, je peux vous le dire, les agriculteurs sont dans beaucoup d'endroits, sur un certain nombre de filières en profondeur, on se cette politique commerciale est d'autant plus reporting Monsieur le Président, qu'au même moment la 1ère économie mondiale, les États-Unis choisi la fermeture et le protectionnisme au même moment, l'OMC n'est hélas plus en situation de faire avancer ses projets au même moment, en revanche, les économies chinoise ou indienne, voient dans le commerce international, un terrain de chasse ou des normes exigeantes et protectrice n'ont guère de place dans le sillage d'une politique commerciale européenne bien conduite, ce sont nos normes sociales, sanitaires, environnementales qui trouveront à s'appliquer, de croire, de croire qu'à terme les citoyens du monde peuvent avoir à y gagner, les normes européennes de devenant en quelque sorte, norme mondiale merci. La parole est à madame Anne-Marie Bertrand, rapporteur de la commission des affaires économiques pour 10 minutes.

Et qui a été adopté à l'unanimité. Aidé par la commission des affaires européennes le 18 janvier dernier est à la fois aux porteurs complet et pertinent, le président de notre commission des affaires européennes Monsieur Bizet en a rappelé le contexte, les enjeux et les principales dispositions. Je m'associe aux remarques qui viennent de formuler j'ajoute qu'au stade de l'examen en commission La commission des affaires économiques, elle aussi, largement approuvé cette proposition de Roger résolution après lui avoir apporté 322. Notre Notre commission a tout d'abord introduit une référence à la notion d'enveloppe globale pour les produits sensibles, je rappelle qu'il s'agit là d'une demande forte des autorités françaises et des milieux agricoles, elle vise à prendre en compte les impacts cumulés des accords commerciaux, à la fois des accords déjà conclus. Et ce, en cours de négociation avant toute ouverture supplémentaire au commerce des filières cible. En effet, seule une prise en compte globale de l'ensemble des contingents d'importations autorisées ou en cours d'autorisation peut permettre de juger si l'ouverture de contingent supplémentaire sera soutenable pour les marchés sensibles comme ceux de l'élevage ou des sucres spéciaux. La commission des affaires économiques, a également adopté l'amendement de notre collègue Marc demandant que soient réalisés des évaluations ex hanté par filière en fournissant une appréciation de nombres d'emplois créés et détruits à court, à court, moyen et long terme. Enfin, la commission a souhaité donner plus de poids à la disposition, qui recommande la mise en place. 2 mesures de sauvegarde pour protéger les filières sensible en indiquant que ces mesures doivent être nos seulement spécifique mais également précise et opérationnelle. Lors de l'examen du texte en commission, j'ai pu percevoir malgré tout quelques interrogations et réticents à soutenir cette proposition de résolution. plusieurs amendements que nous examinerons. Tout à l'heure, exprime ses réserves, je peux les comprendre, même si je ne partage pas toute la politique commerciale de l'Union européenne est un sujet sensible, elle fait depuis plusieurs années l'objet de vives critiques portant à la fois sur les objectifs et le contenu des accords commerciaux conclus mais également sur les méthodes de travail de la Commission européenne. Manque de transparence, manque de réciprocité, manque de réalisme pour ne pas dire naïveté ou encore traitement inadéquat des injures agricole, ce sont les défauts fréquemment dénoncés ici au Sénat, et plus largement dans notre pays. La politique commerciale européenne suscite en particulier une inquiétude très forte pour certains de nos territoire métropolitain ou ultramarin. Et pour certaines de nos filières s'agricoles sensibles tels que la viande ovine et Pauline, le lait et les sucres spéciaux. Une Exposition Sam précaution au commerce international peut mettre ces filières, cela cela tient à différentes raisons et notamment au fait que les normes sanitaires et phytosanitaires sociales et environnementales qui s'impose chez nous sont beaucoup plus strictes que chez la plupart de nos concurrents. Mais c'est bien parce que ces risques sont réels, que la France doit chercher à peser par tous les moyens possibles sur la définition des mandats de négociation des futurs accords et sur le déroulement des négociations. C'est bien parce que ces risques sont réels, qui était important pour nous de soutenir des propositions de résolution pragmatique comme celle que nous examinons ce soir, il peut être tentant de dire que la politique commerciale de l'Europe n'est pas bonne. Elle n'est pas assez protectrice que nous n'en voulons pas de peut-être tentant de dire résident les revend le commerce aux pays qui s'aligne sur toutes nos normes ou excluante purement et simplement les produits agricoles des négociations. C'est un et est-ce que. Que ce de nature à faire. évoluer la politique commerciale de l'Europe d'utiles et bénéfiques pour notre économie et notre agriculture en particulier les accords commerciaux que l'Union négocie prennent en compte les intérêts souvent divergents de l'ensemble des États-membres, la France a ses intérêts offensifs et des fins civiles et elle doit le défendre mais ce qui est bon pour la France, ce n'est pas forcément pour l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne. La réalité c'est que les positions défendues par l'Union dans les négociations commerciales. Sont le fruit de compromis âprement négocié entre les 27 États marbre plutôt que de nouveaux d'du refus de principe confortable ou de soutenir des propositions peu réaliste, il est de notre responsabilité de chercher plutôt à mieux faire partager nos vues. à convaincre nos partenaires par des propositions équilibrées et a pesé sur la définition des mandats de négociation européenne avec des instruments dont nous disposons. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui et l'un de ses instruments, elle reprend nombre de positions défendues unanimement par le Sénat depuis plusieurs années dans des résolutions précédentes, elle reprend aussi plusieurs points de créer du plan d'action relatif à la mise en oeuvre du CETA adopté par le gouvernement de l'année dernière, c'est donc un texte qui contient des propositions à la fois ambitieuse et pragmatique sur les questions agricoles qui sera ça doute au coeur de nos échanges, ce soir, je rappelle que la résolution demande que les produits sensibles, en particulier les produits d'élevage. Ou les sucres spéciaux ou le lait, fasse l'objet de contingent limité demandé qu'il puisse bénéficier de mesures de sauvegarde spécifique effective, elle demandait la mise en place d'un suivi global des contingents à travers la notion d'enveloppe globale ainsi que la reconnaissance du système des indications géographiques. Elle insiste pour que les accords avec l'Australie et la Nouvelle Zélande intègrent dans leur volée développement durable des dispositions contraignantes et opposable dans le cadre des mécanismes inter-étatiques et de règlement des différends. Elle fixe en fait l'objectif d'un degré élevé d'exigences dans l'élaboration de normes communes, sociales, environnementales, ainsi que ça ni. Et phytosanitaire, il me semble que nous ne pouvons que soutenir de telles recommandations. Ne nous y trompons pas, tous les États membres n'ont pas des positions hausse aussi offensive que nous en la matière, il y a un mois, la France qui a souvent été pionnière, a déjà vu plusieurs de ses attentes satisfaite au cours des dernières années, elle doit donc continuer à mettre l'Union européenne sous pression pour faire avancer ses vues, il est utile que le gouvernement qui est en train de discuter avec ses partenaires européens, le texte définitif du mandat de négociation puisse se prévaloir de l'appui du Parlement, cela lui donnera plus de poids, nous devons donc être capable de dégager des positions communes fortes et pragmatique sur des poignets essentiel pour notre pays, gouvernement et Parlement doivent parler d'une seule voix sur ces questions, pour que la France est une chance de convaincre ses partenaires européens. Je voudrais terminer un soulignant quelques enjeux économiques et stratégiques liées à ces 2 accords, la libéralisation des échanges avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ouvrira aux entreprises françaises et européennes de nouvelles au Pérou opportunité commerciale, le commerce de la France avec ces 2 pays est excédentaire, ce n'est plus un cas si fréquemment Jean. Mais nous devons absolument protéger nos filières sensible. Par ailleurs, d'un jeu de ces accords et d'exporter non seulement des biens et des services, mais aussi nos normes sociales et environnementales, ainsi que nos normes en matière de protection des données et de sécurité alimentaire. C'est à nous de peser sur les négociations pour imposer un certain nombre de conditions dans l'accès à notre marché. Nous avons l'opportunité de faire mieux reconnaître certaines de nos noms avec ces 2 accords permettront d'ancrer ces 2 pays dans un système commercial fondé sur des règles alors que le cadre multilatéral se porte mal, c'est peu de le dire, la juge de faire de l'Union européenne, le moteur, le point d'application donne commerciale mondiale, respectueux des règles étonnant jeu stratégique, je vous remercie. Merci, la parole et même. Non Madame Joëlle Garriaud-Maylam, au nom de la commission des Affaires étrangères pour 5 minutes.

nous examinons au travers de cette proposition de résolution européenne les directives de négociations proposée par la Commission en vue d'accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous nous réjouissons bien sûr de la publication de ces directives, qui témoigne des progrès de la transparence mais pourrions-nous nous le demander la transparence suffira-t-elle à obtenir l'adhésion des peuples au projet européen, singulièrement en matière de négociations commerciales internationales et sur le fond, les mandats de négociation proposée par la commission sont-ils de nature à nous rassurer, ils susciteront de ma part 3 remarques tout d'abord sur le périmètre proposé pour les accords, l'objectif prioritaire de la Commission européenne figurant en tête des 2 directives de négociation semble être de restreindre ce périmètre ainsi les accords ne devrait contenir que des dispositions relevant des domaines de compétence exclusive de l'Union européenne, à l'exclusion de tous domaines tous domaines de compétences partagées avec les États membres et donc à l'exclusion de toute ratification des Tursz accord par les parlements nationaux nous approuvons à ce sujet, le texte de la proposition de résolution européenne demandant des négociations concomitantes sur les sujets de compétences partagées et nous nous interrogeons sur l'opportunité d'un découpage en plusieurs accords qui nous conduirait à n'examiner in fine et pour ratification qu'une partie incomplète d'un ensemble dans la logique globale nous échapperait ensuite la transparence cette transparence est un devoir non seulement pour la Commission européenne, mais aussi pour le gouvernement, en amont et en aval des réunions du conseil, mais ce type de négociations internationales et par nature à la main de l'exécutif et peu propice à la publicité. Où peut légitimement s'interroger j'ai sur la portée des informations qui nous sont transmises lorsque l'on apprend, par exemple dans la presse que la commission propose maire sur des quotas d'informer d'importation de boeuf augmenter de 40 pourcent en échange de concessions dans d'autres secteurs sans analyse approfondie de l'impact d'une telle proposition, ce qui donne l'impression que l'on sacrifie les intérêts agricoles européens au profit de ses intérêts industriels, on ne peut pas ensuite cette donnée d'une certaine défiance de l'opinion et d'une certaine perplexité face à la volonté d'ouvrir de nouvelles négociations avec d'autres grands c'est-à-agricole, cela m'amène à mon dernier point, la multiplication des négociations commerciales, la commission est aujourd'hui présente sur tous les fronts, tout en ne délaissant pas les pays s'émergents, elle se tourne aussi vers d'autres pays s'industriel au total une quinzaine d'accords de libre-échange sont en cours de négociation donc fin proche d'un aboutissement avec le Canada, c'est le CETA sur lequel nous devons nous prononcer dans les prochains mois, mais aussi avec le Japon, Singapour, le Vietnam et le maire, tous ces accords sont sensibles quant aux relations avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie 2 accords ont été signés par l'Union européenne avec ces pays, en 2016 et 2017, ce sont des accords mixtes dont nous n'avons pas encore autorisé la ratification, peut-être pourrait-on déjà se donner le temps de les examiner. En conclusion, monsieur le ministre Béchard, collègues, je me demande si la machine n'est pas en train de s'emballer et si la commission Metris vraiment les effets cumulés de tous les accords qu'elle négocie. à ce propos, les dispositions de la proposition de résolution européenne en faveur d'une évaluation renforcée des effets des accords commerciaux et pour une meilleure gestion de Deleuze leur s'impact redistributif me paraissent très je je voudrais, en tout cas, remercié ici ses auteurs de nous permettre de débattre aujourd'hui de ces questions essentielles et remercier également le notre excellent président commission des Affaires européennes, Jean Bizet. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est à vous, Monsieur le Ministre. Bien, monsieur le président, Mesdames et messieurs les présidents, mesdames, la rapporteur mesdames et messieurs, chers collègues, j'allais dire oui reste toujours heureux d'être parmi vous ce soir pour effectivement cette première première je crois effectivement 1er débat sur un mandat de négociation qui n'a pas encore été validé et je crois que c'est tout à l'honneur du Sénat que d'être à l'origine, hé bien de cette initiative et cette application des des parlementaires. Français dès le début du processus de de négociations commerciales qui sont souvent longs ça été rappelé souvent décriés pour leur manque de de transparence et et du coup tout à fait bienvenu et ça va dans le sens des engagements que nous-mêmes nous nous avons pris au gouvernement dans le cadre du plan d'action relatifs au au CETA j', j'y reviendrai un peu alors aujourd'hui je crois qu'on a tout simplement entêté et on le vit aussi sur notre territoire les négociations commerciales font face à une authentique crise de sens et particulièrement en France, on a des concitoyens qui parfois s'interroge sur effectivement, pourquoi la France au travers de l'Union européenne ou de des des négociations avec des partenaires parfois lointain, alors qu'ils éprouvent déjà chaque jour l'impact de la mondialisation économique sur leur vie de tous les jours, parfois de manière positive, mais parfois de manière négative Il était bien que nous ayons le débat aujourd'hui le débat de ce jeu ce soir s'inscrit d'ailleurs dans la lignée d'un certain nombre de débats qui sont tenus dans cet hémicycle, j'en ai le souvenir au moins depuis 2014, mais je crois que Jean Bizet, pourrait nous aider à remonter de quelques années encore, puisqu'il est parti, comment appliquer sur ce sujet-là je salue la une expertise, une expérience chère Sophie Primas n'y voyez pas autre chose, et surtout pas d'impertinence à parce que nous avons à coeur justement nous appuyer sur cette expertise et sa présence d'ailleurs aux côtés du gouvernement à l'OMC en décembre, en atteste

et les élus que que que vous êtes que nous sommes se doivent aussi de pouvoir disposer d'informations plus ample sur le contenu de ces accords et sur l'impact qu'ils peuvent avoir, donc on a, on est face à un enjeu de de légitimité démocratique un ou au niveau national, très clairement lorsqu'on discute, on de ces ces accords commerciaux. En dépit d'un processus de de ratification avec une implication du Parlement européen, on parle souvent, effectivement, de la CGT, avec le, le Canada, le Parlement européen s'est prononcé, c'est ce qui fait d'ailleurs que l'accord a pu entrer en vigueur, de façon provisoire et on est là, on touche à un des fondements de la de la de la de la politique européenne parce que la politique commerciale, si on est bien une dont il a été consenti qu'elle fut transféré à l'échelon communautaire dès le début, c'est bien la politique commerciale et donc à partir du moment où on est authentiquement européen très clairement, le Parlement européen est l'émanation aussi des peuples européens. Et de ce point de vue là le payeur de contestation, néanmoins, nous avons au sein des parlements nationaux, effectivement, notre rôle à jouer et ce rôle je crois il était amené à se développer, justement, de plus en plus en amont, et c'est bien là d'ailleurs, l'exercice que nous conduisons ce soir ce constat, le président de la République l'a établi lors de son discours à la Sorbonne le 26 septembre dernier lorsqu'il a mis l'exigence de la transparence, au coeur des orientations du gouvernement alors. Cette discussion, hé bien est un exemple de bonne pratique et puis nous allons pouvoir évoquer effectivement les objectifs que nous avons les intérêts offensifs que nous défendons et puis les vigilance avoir effectivement sur un certain nombre d'intérêts défensifs.

très régulier auprès des parlementaires sur les positions tenues à Bruxelles et donc ça prend naturellement plusieurs formes : nous sommes à la disposition des commissions compétentes pour répondre sur toutes les questions relatives aux positions françaises lors de l'adoption des mandats et lors des négociations proprement dite, et puis la France s'était engagée dans ce plan d'action c'est à à soutenir la publication des mandats de négociation et d'ailleurs le mandat adopté par le conseil pour le Chili a ainsi été publié en janvier, donc c'est un pas important dans une une bonne direction et puis dans le même sens, la Commission publie maintenant les propositions de mandat, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez le même niveau d'informations que les membres du gouvernement et donc la commission participer elle aussi pleinement à cet effort de transparence. J'ai un souvenir là ils ne sont que transparence se dit aussi Glasnost on va espérer que ça ne se termine pas de la même façon, mais en tous les cas, il est important maintenant qu'effectivement la publication de ses propositions de textes sur le site internet de la commission soit accessible et puis il y a au-delà de la publication des textes bruts, les études d'impact effectivement qui contribue à cette nécessaire je vois d'ailleurs que la commission vous le signaliez Madame la le rapporteur adopter un amendement qui souhaite effectivement le développement de ces études d'impact ex-santé de façon assez détaillée, pour que l'on sache effectivement où l'on va, ajoute que le 2ème amendement significatif que la commission adoptées relatif justement à à l'évaluation dans plafond finalement globale des concessions qui pourraient être consentis par filière sensible est également un amendement bienvenue et ça va tout à fait de position que nous défendons à Bruxelles au quotidien et donc je salue le travail dans c'est déjà fait par la commission avant même que la résolution viennent dans l'hémicycle. Alors s'agissant justement de de l'Australie et la Nouvelle-Zélande il y a aussi une étude d'impact réalisée par la la Commission européenne et menée par la London School of Economics, ce qui prend en compte justement un certain nombre d'éléments économiques, sociaux, environnementaux, donc très clairement on est voilà on s'inscrit de plus en plus je crois dans cette hygiène de vie qui est plus positive, où il y a à la fois la transparence à la fois la, la mise sur la table un certain nombre de données chiffrées et c'est d'autant plus indispensable que le contexte institutionnel de la politique commerciale, il évolue le président Bizet là tout à fait rappelé avec justesse, on a tous en tête les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice d'Union européenne sur le projet d'accord entre l'Union européenne, Singapour qui établit qu'effectivement selon les les stipulations relative à la protection des investissements relevait de la compétence nationale des États et donc prenant acte de cette décision, les 2 projets de mandat, Australie, Nouvelle-Zélande ne comprennent que des éléments relatifs à cette compétence exclusive, alors il y a un débat qui existe d'ailleurs au niveau du conseil voilà les les différents gouvernements États-membres, les discussions sont en cours pour tirer les enseignements de cette décision et très clairement, pour l'instant, on est sur une logique du cas par cas, c'est-à-dire que, il y a pas de

éventuellement remettre en cause tout ce travail patient et bien pose un problème de crédibilité pour l'Union vis-à-vis de ses partenaires et inversement, c'est vrai que ce qui peut plaider pour la mixité, c'est à la fois le fait que nous avons des intérêts offensifs en matière d'investissements qui sont d'autant mieux défendu qu'ils sont partis, qui sont dans la corbeille de l'ensemble des négociations et que, en contrepartie, effectivement, de, de, de concessions commerciales, nous pouvons obtenir un certain nombre de choses en matière d'investissement et de protection nos investissements et puis il y a ce ce ce sujet démocratique effectivement qui permet aux parlements nationaux, de s'exprimer, donc c'est un un débat qui n'est pas un petit débat pour l'instant n'est pas tranché endoctrine je dirais et pour l'instant, c'est une approche pragmatique, je crois qu'il est bien inspire les les États-membres. S'agissant des objectifs des négociations commerciales en question, Australie et Nouvelle-Zélande tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler en 1er lieu que la France, elle est une puissance du Pacifique, je crois qu'on est un certain nombre sur tous les bancs, gouvernement comme comme Sénat hé bien être attaché au fait que la France est un pays du monde présent sur de nombreux continents avec une zone maritime de grande importance et donc cette zone géographique ne nous et donc pas étrangère, et de ce point de vue-là les collectivités d'outre-mer qui constituent une richesse de la France et l'envoi d'éminents représentants ici et cela fait aussi que, hé bien nous avons un certain nombre d'intérêts dans ces zones et notamment cette zone pacifique, nous avons aussi avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des valeurs et des intérêts communs, ce sont 2, démocratie, héritière de la tradition européenne des lumières avec des économies fondées sur la règle de droit à la transparence des procédures, cela ne peut pas nous laisser indifférents, comment dire, en dernier lieu, l'Australie est un partenaire stratégique majeur pour la France, il y a presque un an en mars 2017 les mises, affaires étrangères français son homologue endossé conjointement un partenariat stratégique qui repose sur l'analyse que nous faisons des

hé bien, était en cours d'examen au Conseil d'État, donc cela ne serait tarder mais c'est la vertu de ces débats que pouvoir vous apporter des précisions et des éclairages et puis cette proximité de vues entre l'Union européenne, l'Australie, Nouvelle-Zélande s'exprime aussi dans le domaine commercial, ce sont 2 pays très attaché à une mondialisation régulée par le droit, garantissant une concurrence équitable entre toutes les entreprises, donc il s'agit pas ici de faire des des grandes déclarations de principe, mais de se confronter à une réalité, c'est que le le multilatéralisme commercial traverse une crise profonde.

enfin quand même une faillite à se rendent compte qu'on n'arrive pas à se mettent d'accord pour prendre des mesures et des sanctions contre la pêche illégale la subvention à la pêche illégale, c'est quand même, je trouve assez à Uri sont Vous savez, il y a un certain nombre de critiques qui sont à adresser à ce système multilatéral commercial, les États-Unis sont très critiques vis-à-vis de de l'ouverture commerciale et et considère que les mesures il Natural pourrait frapper directement ou indirectement des intérêts commerciaux de par le monde, nous, nous estimons qu'il faut bien garder une enceinte un forum dans lequel on peut régler les sujets, avoir un organisme de règlement des différends qui fonctionne et c'est vrai que c'est une différence, nous pouvons avoir un certain nombre de rejoint d'un certain nombre de critiques faites par les États-Unis sur les dysfonctionnements du système commercial international parce qu'effectivement il y a un certain nombre de puissances émergentes qui, parfois, hé bien ont tendance à prendre les règles du jeu avec une souplesse, voilà qui est parfois déconcertante et donc nous ne devons-nous pas être naïf et nous adapter à cette, à cette nouvelle donne. Mais en tous les cas, nous avons l'Australie, la Nouvelle-Zélande à bord avec nous pour essayer d'y d'y remédier et donc face au retrait des États-Unis dans une zone marquée par l'émergence forte de la Chine, ces projets d'accords commerciaux très clairement constitue une opportunité pour l'Union européenne et la France pour peser sur les grands équilibres commerciaux du Pacifique, je vous rappelle, c'est une zone quand on regarde l'Australie Nouvelle-Zélande qui vraiment au sud de la zone Asean et puis de la zone Chine-Japon ce sont, c'est là que la croissance mondiale vraiment accélère, hein, et donc c'est là aussi nos entreprises françaises exportent ont un dynamisme de leurs exportations, avons, nous sommes fondés à vouloir, hé bien il pesait plus encore et puis ça a été dit par le président de la commission des affaires européennes, il s'agit aussi à travers ces accords finalement de fixer les normes qui seront celles des produits et services au XXIe siècle, et donc c'est pas une petite affaire, c'est une opportunité aussi historique que de pouvoir faire en sorte que un certain nombre de normes de valeurs européennes et bien dépasse notre continent pour trouver une application ou ou en tous les cas entraîner un certain nombre de partenaires. Alors peut-être quelques éléments complémentaires effectivement sur le contenu de ces projets d'accord avec l'Australie et Nouvelle-Zélande donc depuis la publication des propositions demande à la France négocie au Conseil pour renforcer la partie qui définira les règles des 2 accords commerciaux et donc, naturellement, nous souhaitons que ces accords fasse explicitement référence au respect de l'accord de Paris, c'est d'ailleurs une position que nous défendons. De façon générale, ce qui fait que moi, j'ai souvenir de débattre, nous avons ici dans cet hémicycle, au sujet du projet de traité entre Union pleine et les États-Unis six désuni quitte définitivement l'accord de Paris avec cette règle que nous souhaitons, pas d'accord de Paris égal traité commercial, donc voilà, amis et alliés sont avertis sont prévenus : cette ambition environnementale qui a été je dirais endossée par voilà les États du monde entier, hé bien doit trouver à s'appliquer. Et puis, la France souhaite aussi que les mandats de négociation fasse référence aux conventions de l'Organisation du travail, comment pris position pour que les mandats mentionne dans un autre candidat explicitement le principe de précaution pour qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il continue à s'appliquer sur le territoire de l'Union européenne et puis toujours en cohérence et en application du plan d'actions sur le CETA, la France soutient des amendements aux 2 projets de mandat pour établir Ania explicite entre les accords commerciaux à venir et les travaux en cours au sein des organisations relatives au transport aérien et au transport maritime, et même si l'impact de ces désaccords sur les émissions de gaz à effet de serre du transport international sera réduit, nous devons prendre en compte et réduire cet impact le plus tôt possible en intégrant ces secteurs dans l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de façon plus générale, la France est mobilisée pour que le mandat de négociation incluent une prise en compte transversal des enjeux du développement durable, notamment pour les investissements et les marchés publics, donc vous le voyez, cette politique commerciale, nous souhaitons faire en sorte qu'elles permettent aussi de faire avancer les politiques climatiques et qu'elle permettent mais voilà d'devant une mondialisation régulée, avec un certain nombre de de règles non pas la loi de la jungle et ses enjeux sont donc fondamentaux aussi fondamentaux qui soit, ils ne doivent pas nous occuper occulter le fait que, on a un certain nombre de sujets commerciaux classiques et que ces négociations, ça sera aussi l'occasion de promouvoir des intérêts offensifs et d'être vigilants sur un certain nombre d'intérêts défensifs alors les intérêts offensifs revenons aussi quelques instants c'est naturellement la levée de barrières non tarifaires pour le secteur agricole ou de l'industrie ou l'accès au au marché des services des marchés publics, mais par exemple si on prend le monde agricole avec la reconnaissance et la production et la protection, pardon, des Le CETA a permis la reconnaissance d'un certain nombre d'IGP et JP française ce qui était une première et je peux vous dire, c'est une première qui n'a pas forcément satisfait le grand voisin américain

ces accords permettront également d'éliminer des droits de douane existant dans le secteur industriel et dans secteur agro-alimentaire de manière très concrète en reprenant l'étude d'impact vous en avez parlé, l'accord pourrait ainsi permettre une hausse jusqu'à 27 pourcent des exportations pour la pharmacie, les cosmétiques et le secteur de la mécanique de façon voir ses exportations croître de 63 de même pour les uns, spiritueux de de plus 6 pourcent et pour les fromages de de plus 30 pourcent donc je crois qu'un certain nombre de nos territoires effectivement peuvent y trouver là des raisons d'espérer, mais je vous rassure le gouvernement mesure pleinement aussi la sensibilité de ces de négociations pour les filières agricoles françaises, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont de longue date des exportateurs importants de produits agricoles, du fait de l'Avantage comparatif que leur procure la géographie, donc on a en tête, naturellement, la filière bovine, les produits laitiers, le sucre et les céréales et donc de ce point de vue là la position du Vernon, elle est claire et le président de la République l'a récemment rappelé lors de ses voeux au monde agricole, la France n'acceptera pas que les négociations commerciales conduisent à déstabiliser l'équilibre économique des filières dont nous connaissons la fragilité. Et de ce point de vue là vous savez au mois décembre il y avait des craintes qui est exprimée par la filière bovine par exemple sur la conclusion du projet d'accord soit hé bien qu'il s'est passé au mois décembre à la France avait pas rester les bras ballants, elle a réactivé une coalition de 11 États-membres qui ont des sensibilités agricole, hé bien nous avons pesé, allons peser auprès du commissaire au GAN auprès de la commissaire même Streum auprès des négociateurs européens pour que ces sensibilités soient prises en compte et donc, je peux vous dire que c'est un nous avons cette fois en notre agriculture chevillée au corps et que nous ne sommes pas là pour la braderie très clairement. Et je dis les choses parce que on peut avoir le sentiment dans les prises de parole ici ou là, que la France serait un peu en arrière de la main ma pour être en première ligne sur ce sujet-là, je peux vous dire que, il n'en est rien. Alors il y a très clair que, du coup, le montant des concessions qui pourraient être faites à l'Australie et Nouvelle-Zélande dans ces filières sensible dépendra directement de ce qui aurait pu être concédés au préalable à la fois au niveau de l'OMC 2 avec le Canada, on a en tête les éléments et éventuellement avec le Mercantour parce qu'effectivement on ne peut pas avoir un dit finalement je dirais au fur à mesure que les accords s'empilent des concessions qui s'empilent restant limite et de ce point de vue là ce passage saluer l'amendement de de la Commission sur le plafond des concessions et et sur l'enveloppe globale par filière, que la France défend au niveau européen pour faire en sorte qu'il y ait une visibilité une prévisibilité pour les filières et que hé bien donc voilà trouver leurs équilibres et et avoir en tête le contexte dans lequel vont se se mouvoir et puis nous sommes naturellement toujours à l'offensive pour nous battre afin de mettre en place des clauses de sauvegarde d'étaler naturellement les l'entrée en vigueur d'un certain nombre de contingents et par conséquent je crois que il y a tout un travail d'accompagnement qui qui doit se faire,

des enveloppes qui ont pu être consentis par le passé, parce que sinon effectivement ça peut déstabiliser, enfin, la France sera attentive aux effets éventuels de ces accords sur sur l'outre-mer et notamment sur la Nouvelle-Calédonie, dont l'Australie et la 3ème destination à l'exportation, comme cela était le cas pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre de la négociation, hé bien, de la CGC ta avec le Canada donc au total, nous nous félicitons de la tenue du de ce débat ce soir sur ces 2 projets de 2 mandats de négociation le gouvernement continue à rester à disposition du Parlement dans le cadre constitutionnel pour rendre compte de son action moi d'une équipe d'avoir été un peu long mais j'espère avoir pu vous apporter quelques éléments sur voilà la volonté, la détermination du gouvernement à la fois apporter une ambition au niveau international, au niveau du du du commerce parce que il y a un moment français et ce moment français, hé bien il faut pas le gâcher, il faut l'utiliser à plein, nous nous plaignons parfois de ne pas exporter assez hé bien ces accords de libre-échange sont l'occasion de trouver de nouveaux débouchés, et j'en veux pour preuve. Un rapport intéressant qui a été fait par la Commission européenne justement sur le suivi des accords de libre-échange depuis 2010 et ce rapport a été mis sur la table au mois décembre il indique par exemple sur la Corée, accord de libre-échange qui était, qui est entré en vigueur, provisoirement 2011 définitivement en 2015 et bien que il a permis d'inverser la tendance, c'est-à-dire que nous étions, tenez-vous bien, un déficit de mémoire de lors de 11 milliards d'euros dans le commerce entre l'Union européenne et la Corée, on est passé un excédent de 4 milliards d'euros, donc on voit bien que c'est aussi l'occasion de marquer des points sur des zones qui sont très dynamiques et on aurait bien tort de s'en priver, voilà, Mesdames et messieurs les les sénateurs, quelques éléments sur hé bien ces ces négociations importantes je mesure hé bien la pédagogie qu'il faut faire et c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu long parce que, en fait, hein, nous sommes bien plus nombreuses que ce que nous sommes ce soir dans l'hémicycle ce que dire, c'est que je suis persuadé qu'un certain nombre

le 6 mars prochain hé bien qui sera l'occasion là aussi de faire un point avec toutes les parties prenantes, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Fabien Gay.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues. On aurait compris, j'aurai moi louange sur le libre échangisme que Monsieur le Ministre, mais nous sommes là pour débattre, il y a un an jour pour jour, nous dénoncions l'adoption du CETA au Parlement européen, ce traité véritable cheval de Troie allait ouvrir une voie royale à une nouvelle génération de traités commerciaux qui nie les souverainetés nationales et dessaisit les gouvernements et les parlements de leur libre administration dans l'intérêt général, par des dispositions d'arbitrage de coopération réglementaire ou encore de libéralisation des services et d'ouverture des marchés publics, une vérité éclater au grand jour à traverser divers traités discuter dans un obscurantisme le plus total. Capitalisme libre échangiste est à l'oeuvre dans la quasi-totalité du monde se traduisant par un dumping social et fiscal consistant pour les propriétaires du capital à produire là où le travail est au prix le plus bas et à placer, voire à cacher l'argent là où il est le plus rentable et le moins taxés, tout cela au détriment des peuples pour servir uniquement les puissances de l'argent depuis 13 têtes traité de libre-échange sont en discussion, nous voici donc à discuter, celui qui concerne la Nouvelle-Zélande et l'Australie, 2 poids lourds de l'agriculture extensive et de l'export de viande rouge et de produits laitiers qui ne consomme qu'une petite de leur production, multipliant ainsi les accords commerciaux ambitieux pour développer ce que et sécuriser leurs débouchés de la production australienne est ainsi exporter les réglementations encadrant les filières animales il diffère des exigences européennes, l'utilisation d'hormones de croissance et la décontamination chimique des carcasses, ils sont ainsi autorisés bien que les produits destinés à l'Union européenne ne doit avoir vont revenir au cours ni à Alain ni à l'autre, la traçabilité individuelle et les temps de transport des animaux, ils sont moins strictes qu'en Europe nous couronnes donc double risque que cette règle ne soit ni respectée ni contrôlable, ajoutant que si les opportunités sur ces marchés restent limités pour l'export, les risques sont évidents pour les lots français encore d'octroi d'accès supplémentaire au marché européen, dès lors, du fait de ce déséquilibre, les négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne peuvent pas être considéré comme un partenariat car comment oublier que le secteur de l'élevage et de la production laitière sont déjà en crise dans l'Union européenne et comment ne pas souligner que, du fait des importations de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Notre production ovine peut être totalement démantelée alors que nous la vendent même pas encore réglé les différends à l'OMC sur la répartition des constats d'importations agricoles qui découle du Brexit, voilà que nous négocions avec 2 géants agricoles parmi les plus compétitifs au monde alors que tous les contingents tarifaires qui pourraient être accordées à ces pays auront vocation à l'issue du Brexit à s'impliquer un marché communautaire réduit alors que, comme cela a été très justement rappelé lors des débats en commission, les états généraux de l'alimentation viennent à peine de s'achever et qu'un projet de loi nous sera prochainement présenté comme l'a justement dit mon collègue milliers il sera en totale contradiction avec les accords d'Oslo nous débattons, on ne peut pas demander toujours plus de normes pour nos produits et ouvrir largement notre pays a des aliments qui ne respectent pas les contraintes que nous impose dès lors poursuivre ces négociations après le CETA et la volonté affichée de la Commission, de lancer un autre traité avec le maire pour sourds, c'est signé la mort d'une agriculture paysanne, garante d'une alimentation de qualité et de l'emploi, or et ce point est essentiel tôt dans un accord de libre-échange relève de la compétence exclusive de la Commission européenne, sauf le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États cette position a été rappelé par la Cour de justice, dans un avis du 16 mai 2017 en conséquence après conclusion de l'accord et aval du Conseil et du Parlement européen, les parlements nationaux ne seront pas concernés c'est l'également le cas de la elle avait le Japon qui a été finalisée à la fin de l'année dernière, enfin, le Conseil ne devra plus se prononcer sur l'accord final, à l'unanimité mais à la majorité qualifiée ainsi les États sont doublement exclus du processus décisionnel et ce déficit démocratique de l'Union européenne n'est pas acceptable au vu des enjeux que comporte de tels accords désormais d'une agriculture paysanne locale de taille humaine et respectueuse de l'environnement que l'on va sacrifier pour lier notre alimentation aux chaînes de production mondialisés de l'agro-Business là où nous disposions de viande de qualité produite localement avec la meilleure traçabilité nous allons-nous léguer avec les producteurs à des milliers de km, c'est d'ailleurs le sens de nos amendements sur la préservation de l'eau de la ruralité et de l'accord des parlements nationaux, certes la proposition dont résolution dont nous débattons aujourd'hui va dans le bon sens en cohérence avec les différentes positions du Sénat en la matière, et en particulier des propositions que notre groupe apporté, certes il faut plus de transparence et n'aurait réciprocité certes, il est nécessaire que les futurs elle plus un volet environnemental et social opposable certes nous souscrivons pleinement la nécessité que les produits d'élevage et les sucres spéciaux nie s'être l'objet de contingent limité un n'allemande des période de démantèlement tarifaire et que soient prévues des mesures de sauvegarde spécifique mobilisable rapidement en cas de déstabilisation des filières concernées sous l'effet des importations toutefois face à des accords aussi importants, les parlements nationaux doivent être saisies au fin des ratifications pour conclure : nous pensons que les produits sensibles doivent purement et simplement être exclus du Champ de la négociation, fondamentalement, la multiplication des accords de libre-échange, alors que les difficultés structurelles de notre agriculture n'ont pas été Rosol et tu fuite en avant mortifère, c'est pourquoi nous ne voterons pas l'État pour cette proposition de résolution qui ne fait que accompagner un mouvement de mise en concurrence que nous dénonçons et que continuerons rendent continueront à dénoncer de manière systématique sur les blancs de cette assemblée,

Monsieur le président, Monsieur le ministre, mais cette dame, messieurs les rapporteurs mesdames messieurs. J'aurais vous l'imaginez, au nom du groupe centriste. Un discours quelque peu différent de ce qu'on vient d'entendre, tout simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, ni la France ni l'Europe ne ne peuvent être renfermée sur elle-même. On n'est pas forcément d'accord sur un libre échange intégral et totale, mais je crois qu'aujourd'hui il y a des intérêts communs à signé des accords avec un certain nombres de pays à travers le monde surtout à un moment où les États-Unis se renferment sur eux-mêmes et veulent être les capitalistes du monde mais non plus les économistes du monde. Je crois qu'aujourd'hui l'intérêt de la France clair à travers l'océan Pacifique, la Nouvelle Calédonie, qui se trouve à proximité et la 3ème, île du Pacifique et que nous avons intérêt à entretenir des échanges, mais des échanges qui ne sont pas tout à fait nouveau, il y a bien longtemps que le mouton de Nouvelle-Zélande est venu sur le marché européen que la laine de Nouvelle-Zélande est devenue sur le marché européen certes en fragilisant une agriculture certes en fragilisant une économie et c'est vrai que pour l'agriculture, c'est un choc de civilisations entre je dirais l'agriculture du Nouveau Monde et l'agriculture, des des vieux pays du continent européen, mais je crois que. Notre pays, l'Europe toute entière peut défendre l'intérêt de son économie peut défendre dès les accords de libre-échange. Tout en étant fermes dans les négociations. Je crois que le risque aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'agriculture française est en crise, ça n'aura échappé à personne. Je le rappelle souvent un Pierre des agriculteurs gagnent moins la moitié du SMIC et qu'aujourd'hui ils sont inquiets pour leur et agriculture et que l'Europe doit non seulement les rassurer mais elle doit les protéger. Je crois que nous. Fonctionnaires et parlementaires européens ont encore une vision un peu trop peu Angélique d'une politique libérale et libre échange j'étais voilà quelques jours, au Canada, où on vient de signer des accords de libre-échange, hé bien les producteurs laitiers voient leur lait payé 1 Pierre plus cher qu'en Europe. Ils ont des accords de libre échange avec l'Europe, et en même temps ils savent protéger un élevage laitier au Canada et je crois que aujourd'hui. L'Europe doit comprendre qu'on peut être libéral, on peut avoir des partenaires économiques dans le monde, mais que l'Europe ne doit pas être en quelque sorte la passoire. L'Europe a été établi un certain nombre de normes de production pour les produits et pour les consommateurs européens, tout simplement en mettant en avant la santé publique en mettant en avant l'environnement de notre pays. En démontrant aux agriculteurs que leur avenir passait par des efforts importants sur la qualité sur la diminution des pesticides sur la fin, sur une production animale sont hormones sans antibiotiques. Et je crois qu'effectivement il n'est pas possible d'expliquer aux agriculteurs français et européens que des accords de libre échange ne doivent parce appuyée sur des contraintes concernant les produits importés. Je crois que les produits importés qui viennent en Europe doivent respecter les mêmes règles, je dirais, de production, comment imaginer que les feux français ou européen élevé sur un parcours en herbe et doivent être produits au même prix que des vieux produits dans des Budgets in dans des cages de poules pondeuses en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tout simplement, il y a Béziers règles et des normes de sagesse l'Europe attend des produits de qualité, nous ne pouvons pas laisser entrer n'importe quoi sur le marché, même si au niveau des OGM, l'Australie, protège et n'a pas pris le parti de produire des céréales avec OGM, l'agriculture de ces pays là et l'élevage notamment utilisent très largement ces produits qui ne sont pas autorisés en Europe et je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai débat de compétitivité notre agriculture peut-être compétitive si on lui fixe des règles de concurrence loyale. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, l'Europe doit prendre sa place dans le monde, y compris à travers des corps commerciaux mais en même temps l'Europe doivent être un exemple doit être un exemple en matière environnementale, à travers des règles de production, c'est vrai que quand on connaît par exemple les règles sanitaires pour l'élevage et l'agriculture française ou européenne, quand on connaît les conditions d'élevage. Allez voir des bovins d'engraissement dans ces pays, nouveau, et bien je puis vous dire que les normes environnementales et l'énorme pour le cheptel n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous, hé bien sûr, lorsqu'on a Libre-échange : il faut avoir des agriculture compétitive, il faut être capable de supporter la concurrence ou alors il faut être capable d'imposer des règles que l'Europe a fut imposée, a fait 20 agriculteurs et qui protège les consommateurs et je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement le défi est-ce que l'Europe en négociant des traités de libre-échange est capable en même temps d'avoir de l'ambition pour son agriculture et pour son économie toute entière, donc aujourd'hui c'est le vrai défi, l'Europe ne doit pas avoir une guerre de retard, l'Europe doit s'ouvrir sur le monde et en même temps, l'Europe doit comprendre qu'une économie ça se protège et que pour cela à travers les négociations je suis surpris de voir qu'on en voit beaucoup trop facilement des commissaires ou des hauts fonctionnaires européens pour négocier, je prends l'exemple du Canada l'ambassadrice du Canada était une chef d'entreprise qui s'est mis en disponibilité pendant 5 ans pour prendre un poste d'ambassadeur et bien sûr pour faire comprendre que les traités de libre-échange avec le Canada peuvent être négociée et discutée avec la France et avec l'Europe et je crois que demain il faut que dans ces négociations, il y a, je dirais un peu plus de tempérament anglo-saxon et ce tempérament, on le perd un peu avec le départ des Anglais parce que on pense que le libre-échange, c'est d'ouvrir les portes et de ne rien négocier, moi je ne suis pas favorable à des quotas qui protégerait et qui n'apporte forcément pas grand-chose, mais par contre je crois que les règles imposées par l'Europe à ses producteurs doivent s'imposer de la même monnaie, manière aux produits qui feront importée en France et en Europe.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, j'associe l'intervention mon collègue Marc Denis, ce qui est retenu en circonscription. L'examen aujourd'hui de 2 projets de mandat de nouvelle génération de nouvelles négociations commerciales entre l'Union européenne et respectivement l'Australie et la Nouvelle-Zélande est le fruit d'une victoire dont nous pouvons nous féliciter nous féliciter d'exercer un droit acquis de haute lutte, grâce au combat mené par la France de l'adoption du mandat sur la négociation pour un partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis est poursuivi lors de la phase finale de l'accord CETA conclu avec le Canada, les parlementaires de tous les États membres peuvent désormais officiellement s'exprimer sur le projet de mandat de négociation commerciale que la Commission européenne propose d'engager au nom de l'Union européenne avec d'une part, l'Australie et d'autre part, la Nouvelle-Zélande. Il y a un intérêt stratégique à développer ses partenariats si l'Union européenne n'y va pas, c'est avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud, que l'Australie, la Nouvelle-Zélande développeront leurs échanges selon des règles et des normes que nous ne maîtrisons pas et qui pourrait, si on n'y prend pas garde, s'imposer à nous par la suite, les parlementaires ont également gagné ces dernières années un droit de suivi des négociations, grâce notamment à la mise en place d'un comité stratégique de suivi des négociations commerciales qui fonctionne bien, mais les parlementaires dans le même temps, ont perdu le droit de voter, à postériori, ces accords. Et ça, nous pouvons effectivement le regretter. Cette implication progressive des parlementaires est essentiel, alors que la Cour de justice de l'Union européenne dans son avis sur l'accord, Union européenne, Singapour a conforté la Commission européenne dans sa compétence est-ce en matière de négociations commerciales je voudrais toutefois souligner ici que la question de la conclusion d'accords de libre-échange relevant uniquement de la compétence exclusive de la Commission européenne fait toujours débat et n'a toujours pas été tranché, la Commission européenne s'est pour l'instant, engagé à ce que cette compétence exclusive ne soit pas automatique. Ses premières expériences de contrôler suivi nous permettent aujourd'hui de mieux anticiper et défendre les intérêts européens et nationaux, d'être mieux armés sur la scène commerciale internationale mais aussi d'entrer plus sereinement dans le débat démocratique en même temps, nous devons absolument répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, elles sont légitimes, la première réponse et la grande transparence et le renforcement du contrôle démocratique sur ces négociations commerciales, mais nous devons, allons plus loin, plus loin encore, nous devons assurer un véritable équilibre entre protection et ouverture et ce pourquoi nous nous battons depuis des années et notamment au Sénat. L'expérience des dernières négociations commerciales vient conforter cette position cette conviction qu'il faut continuer à se battre à promouvoir notre modèle de développement que tirer en réalité de l'échec des négociations du thé, c'est qu'à un moment donné, un État membre, comme la France peut dire qu'il n'y a pas assez d'avancer pour faire des concessions supplémentaires et que l'Union européenne ne peut pas aller plus loin, que dire de la réouverture in-extremis de la négociation de l'accord CETA. C'est que lorsque porte des propositions légitime, on peut peser et même réformer, faire évoluer les mentalités, sans cette conviction, nous n'aurions pas un mécanisme d'arbitrage qui puisse préserver le droit et réguler les États-membres et protégés dans les recoins par des recours, nous n'aurions pas ses exigences développé dans cette proposition de résolution européenne. Alors nous repliant par l'Union européenne a les moyens et la responsabilité de peser sur les normes Euro commercial international, c'est d'ailleurs le bilan des débats dans nos commissions respective, il faut aller plus loin dans le de nos exigences pour l'Union européenne puisse aborder les négociations commerciales en défendant au mieux les intérêts européens, ceux des citoyens, ceux des consommateurs et bien sûr ceux des producteurs. Ces accords de nouvelle génération ne sont plus seulement des accords commerciaux mais des accords qui doivent nous permettent de défend des valeurs défendre un modèle de régulation commerciale et de border des mandats de négociation. Nous saluons les propositions de ces peuples, s'être cet air comme l'exigence de transparence de l'ensemble du processus de négociation et nous comptons bien que le gouvernement nous rendent régulièrement compte de son avancée comme le caractère contraignant et opposable des dispositions communes en matière de développement durable environnemental et social, ce qui constituerait une avancée majeure, s'il était validé. Nous voudrions ajouté que toutes ces demandes, constitue pour nous une ligne rouge, il faudrait au niveau européen, aller plus loin, un travail de l'évaluation en amont des négociations afin d'anticiper et de mieux prévenir les effets économiques et sociaux des accords commerciaux. Notre principale préoccupation pour cette PPR a été de travailler à l'anticipation et la prévention des compétences négatifs de l'ouverture de nos marchés plutôt que de seulement tenté de les réparer, je crois que la Commission européenne n'a pas assez travaillé dans ce sens, c'est un travail essentiel qu'elle doit faire et que les États membres doivent soutenir le gouvernement doit faire des propositions en ce sens, c'est le sens de nos amendements que nous porterons tout à l'heure et qui ont reçu un accueil favorable de la en commission des affaires économiques et qui vise notamment à renforcer le poids et les exigences de cette PPR. Nous avons un modèle dans ses négociations commerciales, à nous de savoir les de fondre le pouvoir pour cela tout un travail reste engagé au niveau européen et nous comptons nous parlementaires, il y a être associés et prendre toute notre part merci. Merci donc la parole est maintenant à Madame Colette Mélot. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons cette résolution, dans un contexte politique particulier, tant pour la construction européenne que pour le processus de mondialisation économique que nous connaissons depuis plusieurs décennies en ce qui concerne l'Union européenne, les crises sont connus : crise du Brexit crise démocratique crise migratoire crise morale même je n'y reviendrai pas en ce qui concerne la mondialisation des échanges qui prévaut depuis des années 90, la crise est plus insidieuse remise en question du multilatéralisme par les grandes puissances, mise en place de stratégies commerciales agressives, rejet du libre-échange, nous sommes à un tournant ou le retour du protectionnisme et les blocages de l'Organisation mondiale du commerce, menace un système économique mondial fondé sur la libre circulation des biens, des capitaux et des hommes, la politique commerciale de l'Union européenne est au coeur de cette double crise à la fois, crise de légitimité de l'Union et crise du système économique mondial, nous l'avons vu avec les débats autour du TIP, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, nous l'avons vu les débats autour du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, une crise de légitimité d'abord dû à un déficit de transparence et de démocratie dans la négociation des accords commerciaux, il faut néanmoins se féliciter des mesures prises par la Commission pour remédier à ces critiques depuis quelques mois, par exemple la création d'un groupe consultatif sur les accords commerciaux ainsi que la publication des directives de négociation et des études d'impact sont des pas importants en direction d'une meilleure visibilité de la part des citoyens, nous nous associons à l'appel lancé dans cette résolution pour que la commission accentue son effort de transparence en direction des Parlements nationaux et du gouvernement une crise d'efficacité, d'autre part, dans un contexte de concurrence mondiale ou la naïveté se paye comptant face à des blocs économiques puissants disposant souvent d'arsenaux réglementaire et tarifaires performant, la Commission européenne est souvent accusé de sacrifier les intérêts commerciaux des États-membres. Le principe de réciprocité notamment doit faire partie des lignes directrices, directrice de nos négociations commerciales, en particulier en terme de marchés publics,

Nos concitoyens ne comprennent plus ces différences, il est heureux que le texte de cette résolution rappelle cette exigence. Une crise enfin dans la protection de nos standards élevés en matière environnementale, sociale et culturelle standards élevés font notre fierté et constitue un modèle de société que nous devons promouvoir dans le monde. La Commission européenne doit on doit un être la garante et veiller à ce que les accords commerciaux préserve un niveau de protection important pour nos concitoyens, une Europe qui protège ce n'est pas une Europe protectionniste, c'est une Europe plus juste et plus forte. Nous saluons ainsi le texte de la résolution lorsqu'il demande que les futurs accords incluent un volet environnemental et social opposable aux parti. Nous appuyons les mécanismes de protection de nos éleveurs. Face à la puissance agricole de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes d'accord enfin avec les appels allié de libre-échange et renforcement du Fonds européen d'adaptation à la mondialisation pour protéger les travailleurs les plus fragiles. Je vous proposerai moi même un amendement appelant le futur accord respecté la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles dans les dispositions relatives aux services numériques et au E-commerce. Sous la présidence de Jean-Claude Junker, la Commission européenne a tenu compte de cet enjeu de la maîtrise de de la mondialisation dans ses réflexions. Le modèle européen équilibré entre laisser-faire à outrance et un protectionnisme dangereuse est une chance pour une mondialisation plus juste cette résolution sur les accords commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande et l'opportunité de réaffirmer cet espoir. Pour toutes ces raisons et parce que nous nous battons pour cet espoir d'une Europe plus forte dans un monde plus juste mon groupe, les indépendants républiques et territoires votera en faveur de cette résolution, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des affaires européennes, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteur qui est officier pour la première fois dans ce dans je voudrais saluer la cette proposition de résolution européenne qui nous est soumise aujourd'hui. Et qui nous permet de, de, de débattre de ce sujet d'une haute importance. Ces dernières années, l'Union européenne multiplie les accords de libre échange afin de conforter sa place d'acteur majeur des échanges internationaux les plus récentes des TIP le site la l'accord Mercosur font et ont fait l'actualité ont provoqué aussi une énorme mobilisation de l'opinion publique, ces accords successifs nous pose plusieurs questions à la fois sur les aspects démocratiques de leurs négociations et sur leurs impacts sociaux et environnementaux tout d'abord la compétence exclusive de la Commission et le manque de transparence des négociations post-un problème démocratique, nous sommes aujourd'hui en position d'observateur, car je crains que pour ses accords avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Australie, le Parlement soit privé de ratification parce que ce sont des accords non mixtes, nous proposerons d'ailleurs un amendement pour contester cet abandon sur la question de l'opacité des négociations, rappelons qu'il a fallu à l'occasion du TTP taffetas que l'opinion publique et que les parlementaires nationaux, notamment chez nous sans saisissent et contraignant la Commission à plus de transparence. Sur la question des impacts sociaux et environnementaux nous reprochons à la Commission européenne de ne pas exiger suffisamment de réciprocité de réciprocité des partenaires, en particulier sur les domaines sanitaires et phytosanitaires nous accusons également à la commission de sacrifier certains secteurs pourra tenir un bénéfice global pour l'Union européenne, c'est le cas dans le cadre de chacun d'être traités de ces traités pour les productions agricoles et alimentaires trop souvent considérés comme des valeurs variable d'ajustement, le secteur de la viande bovine déjà extrêmement fragile sera nécessairement déstabilisés par les contingents massifs prévus par les accords du CETA et du Mercosur ce même problème sera encore aggravée par l'accord, qui fait l'objet de nos discussions, pour les secteurs des viandes bovines mais aussi ovine, celui du lait et celui des sucres spéciaux qui concernent nos territoires ultramarins face à ces enjeux, les exigences formulées par ce texte de PPR sont tout à fait pertinente, nous tenons à saluer la demande d'une plus forte transparence. Sur la limitation des impact sociaux et environnementaux, nous sommes favorables à l'exigence d'un volet environnemental et social opposable ainsi qu'aux demandes sur la réciprocité, enfin, le texte propose de protéger les secteurs sensibles, notamment par l'aliment, limitation des contingents pour les produits d'élevage et sucre spéciaux. Saluons ont encore cette initiative de résolution et la qualité des échanges qu'elle a provoqué en tant qu'écologiste. Rattaché au groupe RDSE, j'ai le plaisir d'annoncer une approbation unanime de ce texte par notre groupe, enfin en conclusion mon propos, je voudrais vous dire qu'au fond de moi. Je crois vraiment que ces accords de libre-échange intégrant les productions alimentaires n'iront plus très loin dans leur application, parce que l'on ne va pas pouvoir continuer comme cela, le grand marché international des denrées alimentaires nous conduit au bord du gouffre et est en train de la mine et l'ensemble des produits petits producteurs chez nous comme ailleurs, alors qu'à l'échelle de la planète, un travailleur sur 2 est encore un paysan, je crois vraiment en la le Roeulx relocalisation de l'alimentation, cela dans l'intérêt des paysans d'ici et d'ailleurs dans l'intérêt des territoires des consommateurs de la santé de la biodiversité, nous aurons l'occasion d'en débattre lors de la prochaine loi concernant l'agriculture et l'alimentation des réflexions particulièrement intéressantes sont menées sur cette relocalisation de l'alimentation et aussi, madame la présidente de la commission des et des affaires économiques. Je vous invite à solliciter monsieur Olivier De Schutter. En audition par notre commission cet ancien rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation mène actuellement un travail sur une nouvelle PAC PAC comme Politique alimentaire commune. Et je vous soumettrai également une autre proposition d'audition, celle du cabinet cela groupe pour la présentation de son scénario after 2050 qui définit des trajectoires de transition agricole, alimentaire et climatique qui nous sont nécessaires, je tenais à vous en parler tant le modèle de développement. Annoncée. Personnellement, me donne le blues et me déprime, il est temps de remplacer l'économie de la surabondance par une économie de la résilience pour cela, je fais partie de celles et ceux, de plus en plus nombreuses et nombreux, qui plaide pour une gouvernance mondiale démocratique de l'alimentation, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Monsieur André Gattolin. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je veux me réjouir ici que nous puissions nous prononcer ce soir sur les orientations à donner à aux 2 mandats de négociations en vue d'un accord du Bressan avec d'une part, l'Australie et d'autre part, la Nouvelle-Zélande, je tiens en repère remercier tout particulièrement nos 2 collègues réalisateurs et Marie est à l'origine de cette PPR et au ministre le Moine qui suit avec vigilance et grande ouverture 10 pris ces dossiers si, comme le président de la République et le gouvernement de la France, nous ne cessant de prôner le retour à une approche multilatérale des échanges économiques et pas que des échanges économiques, nous sommes aussi conscients que l'inertie actuelles de l'OMC ne doit pas pousser l'Union européenne à la paralysie, l'Europe doit continuer de s'affirmer comme une puissance économique et utiliser l'existence d'accords bilatéraux de libre-échange comme un levier pour promouvoir des normes européennes ambitieuse tant sur le plan sanitaire environnement peu sur celui qu'on oublie souvent de sites de respect des droits fondamentaux, la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont pour nous des partenaires historiques doté d'institutions démocratiques, avec qui nous ne devons cesser de renforcer nos relations tant pour notre bien réciproque comme pour celui de l'équilibre est de l'ordre mondial ces dernières années, ces 2 pays ont de leur côté, il faut bien le dire, multiplié des accords commerciaux avec d'autres partenaires, la Chine, le Japon, la Corée du Sud sont devenus des fournisseurs et des clients de premières heures pour ces 2 nations récemment, vous le savez, les États-Unis ont renoncé à développer leurs relations commerciales avec la zone Pacifique et pas que la zone Pacifique d'ailleurs plus récemment encore, la décision britannique de quitter l'Union pourrait avoir des conséquences majeures sur les échanges commerciaux importants qui subsistaient, notamment entre le Royaume-Uni et ces 2 membres historiques du Commonwealth, il apporte donc que l'Union européenne puissent maintenir des relations économiques étroites avec ces 2 pays le 1er ministre australien qui était en visite à Londres en juillet dernier a d'ailleurs rappelé que, je le cite, s'il était très désireux naturellement de nouer des accords commerciaux commerciaux avec le Royaume Uni, après sa sortie de l'UE, ils souhaitaient en 1er lieu conclure un accord avec l'Union européenne, de fait, nos pays bénéficient d'une balance commerciale nettement excédentaire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, mais cette situation est loin d'être acquise bouleversements des bouleversements en cours dans le commerce mondial aussi si ces 2 projets d'accord se profile sous des auspices et dans des perspectives qui sont globalement positifs, nous devons cependant être tant tant sur le fond que sur les modalités de négociation à ouvrir, car l'hostilité manifestée par nombre de ses nos concitoyens à l'égard du taffetas et désaccords c'est ou des actuelles négociations avec le Mercosur sous crée un climat de défiance fort à l'endroit de tous les traités en cours de discussion à venir l'Union semble avoir partiellement au moins tirer certaines conséquences d'ailleurs de ce climat, les engagements pris par la Commission dans son nouveau paquet commerce de septembre dernier, sont plutôt encourageants, même s'il mérite certainement d'être encore approfondi, comme d'ailleurs le préconise le texte que nous examinons la véritable transparence devrait être instauré quant au mandat de négociation, confié à la Commission, toutefois, ces négociations doivent être menées avec lucidité et sans naïveté, aussi je me félicite de l'action offensive menée par notre gouvernement à travers son plan d'action pour la mise en eau du CETA qui poussent aujourd'hui la Commission européenne a adopté une posture plus ambitieuses lors des prochaines négociations commerciales en faveur d'une meilleure prise en compte des enjeux sanitaires et de développement durable et ainsi que de lutte en faveur de la préservation du climat, je veux saluer ici l'ambition de notre gouvernement d'intégrer dans les futurs accords commerciaux renvoi explicite à l'accord de Paris et à la coopération dans la lutte contre les changements climatiques. De même, il faut reconnaître que les engagements pris d'associer le Parlement à ses travaux et de le tenir informé tout au long de la côte, vite des noms que négociation commerciale de la part de notre gouvernement, vont dans le bon sens, j'espère seulement que cette volonté sera reprise par les autres États-membres, mais aussi par la Commission comme nos collègues, rapporteur de cette PPE je ne vous cache pas que le groupe la République en marche du Sénat est lui aussi très sensible à la délicate question des secteurs précisément qualifiés de sensible, de nombreuses inquiétudes pointent l'insuffisante prise en compte des impacts négatifs de la libéralisation des échanges, en l'état actuel, les pays de l'Union sont dans une situation de faiblesse compétitive face à la Nouvelle-Zélande et l'Australie dans un certain nombre de secteurs, notamment agricoles, puisque nos filières sont c'est vrai tenus de respecter des exigences environnementales, sanitaires et phytosanitaires et de bien être animal bien plus élevé, l'Australie et notamment à producteur significatif de sucre, tandis que la Nouvelle-Zélande est actuellement le plus grand exportateur de produits laitiers au monde, dès lors qu'il apparaît essentiel de veiller à protéger nos produits agricoles sensibles qu'il s'agisse des filières bovines, ovines ou encore des produits des régions ultrapériphériques dont on particulier les sucres et cette sensibilité doit absolument être pris en compte dès le mandat de négociation à ce sujet et contenu des diverses négociations en cours, nous demandons que l'Union européenne adopte une approche basée sur le cumul des concessions effectuées dans les négociations, c'est avec celles et ceux en passe de l'être dans d'autres négociations à venir produit Cencic par produits sensibles, comparativement à la capacité d'absorption du marché intérieur, une telle approche à la fois cumulative et panoptique serait une partie du remède face à des inquiétudes bien légitimes légitimes donc pour conclure et au-delà de ses points de vigilance et d'examens qui sera réservé aux amendements, le groupe la République en marche, il faudra en faveur de ce texte.

Monsieur le président, Monsieur le ministre, mais chers collègues dans quelques jours, le Conseil de l'Union européenne se prononcera sur les projets de mandat sollicité par la Commission européenne pour entamer la négociation d'accords commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Permettez-moi, en préambule de mon intervention et comme cela a été rappelé par le président Bizet d'autres orateurs même félicité que la commission, elle, pour la première fois accepté de mettre immédiatement ces documents à disposition du public cet engagement en faveur d'une grande transparence était profondément attendu, il était en effet indispensable pour renforcer la légitimité de la politique commerciale européenne de répondre à l'émotion, la défiance, voire la suspicion suscitée chez nos concitoyens par le secret qui entoure d'habitude et négociations commerciales. Ce changement de méthode permet également aux parlements nationaux de se saisir très en amont de ces projets d'accord pour marquer dès le début du processus de négociation certaines exigences fondamentales comme celles qui sont contenues dans la présente résolution je souligne néanmoins que cette effort de transparence devra se poursuivent tout au long des discussions étant donné l'impact potentiel de ces accords sur notre économie et ne territoire il est essentiel qu'à chaque étape, les parlementaires soient tenus pleinement informés par le gouvernement du développement des négociations. Il ne sera d'ailleurs pas moins primordial à l'avenir de contrôler davantage la mise en 9 des exigences en contenues dans ces accords et de surveiller plus étroitement encore leurs impacts économiques cumulées. Mais si nous devons naturellement exercer une vigilance exigeante et Constantin tâchons également de considérer les accords commerciaux pour ceux qui sont, c'est-à-dire des sources d'opportunités, et pas seulement de menaces, rappelons-nous qu'à ce jour, union européenne demeure la principale puissance commerciale au monde. la fois et la France dispose d'atouts tout à fait considérables à faire valoir sur les marchés mondiaux, y compris d'ailleurs dans le secteur agricole et agroalimentaire qui cristallise en tant d'inquiétude. ou pas, que certaines de nos filières sont clairement à l'offensive dans ses négociations et quel bénéfice Ciron grand demande la levée des diverses barrières tarifaires et non tarifaires de nos partenaires, pourvu bien sûr que nos différentes normes ne soit pas battu en brèche. Pour celles qui seront structurellement plus vulnérable à la libéralisation des échanges, des mesures d'encadrement et d'accompagnement sont bien entendu nécessaires, outre la nécessité d'un soutien financier adapté d'un classement en tant que produits sensibles qui doit notamment permettre l'offre de contingents tarifaires aussi limitée que possible, je souhaiterai insister sur la question des clauses de sauvegarde, là où les Italiens une ligne n'hésita généralement pas agi en quelques jours, avec des mesures massives, la mobilisation de ces mêmes clause en Europe souffrent généralement du syndrome du trop peu et trop tard. Cela n'exonère évidemment pas les filières concernées d'une nécessaire réflexion sur leur organisation, leur position sur les marchés et la mise en place de stratégies plus offensive à l'export. Mais si l'Union européenne veut éviter des procès en naïveté commercial qui lui sont régulièrement intenté il est indispensable que la commission évolue dans sa pratique, elle a certes commencé à le faire dans d'autres domaines avec la modernisation bienvenue de nos outils de défense commerciale. Mais il faut désormais que nous soyons extrêmement attentifs à ce qu'elles agissent plus vite et de manière appropriée face aux perturbations des marchés qui pourraient résulter de l'application de ce futur accord comme d'ailleurs de ce qui ont été conclus par le passé. Si nous devons, à l'évidence montrer moins frileux vis-à-vis de la mondialisation, nous ne pouvons pas non plus rester passif face aux dégâts qu'peut également provoquer et ce, alors même que des outils de protection sont à notre disposition. Le refus de la protection légitime mais n'aurait alors inévitablement au protectionnisme qui ne ferait qu'affaiblir l'Europe or dans un contexte international marqué par le recul du multilatéralisme, par l'effacement relatif des États-Unis et la montée en puissance de la Chine, l'Europe ne peut rester en retrait et doit se montrer compte conquérante et offensive en pour s'affirmer comme la grande puissance commerciale qui est. C'est d'autant plus vrai qu'il s'agit de conclure des accords et donc de renforcer nos relations avec des pays qui partagent nos valeurs et nos modes de vie et qui ont donc une vocation à compter parmi nos plus proches alliés dans un monde chaque jour un peu plus incertain, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le ministre, mais cher comme un collègue, comme cela a été dit, nous avons à débattre de la proposition de résolution européenne sur les directives de négociations en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'autre part. Ce texte a vocation à nourrir les négociations de 2 accords disjoints mais cependant concomitants qui vont s'ouvrir avec ces 2 pays, sans exagérer outre mesure l'importance du moment, il convient de le relever, c'est la première fois que le Parlement ait amené à évaluer un mandat de négociation avant que celle-ci soit du moins officiellement, si ce n'est ni sciatique qui fut prise pour le TIPP par notre regretté collègue Nicole Bricq en 2013. Cela renvoie tout d'abord un contexte particulier qu'il faut souligner, car il explique que le 1er point majeur de cette proposition de résolution européenne, nous ne nous prononcerons pas ce soir sur le contenu d'un futur accord de libre-échange, mais bien sûr le mandat que nous entendrons voir accorder à la Commission européenne. En effet, depuis l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne 16 mai 2017, il apparaît que la quasi-totalité d'un accord de libre-échange relève de la compétence exclusive de la Commission. Cela très probablement interrogé certains d'entre nous pour des raisons d'ailleurs d'ailleurs diverses mais en tout état de cause, telle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés l'enjeu éminemment politique de nos débats et donc de déterminer dans quelle mesure nous arriverons malgré ce cadre contraignant à peser sur le contenu d'un éventuel futur accord de libre-échange. Nous avons en la matière, 2 positions possibles, un rejet de cette réalité et par voie de conséquence de ce texte qui nous empêcherait de transmettre à la commission des directives de négociation, l'autre méthode consiste à faire part à la Commission européenne de nos points de vue quant à l'ouverture de ces négociations qui ne vont pas sans poser plusieurs questions : c'est le moment crucial de nous exprimer, parce qu'il s'agira du seul les accords commerciaux ne seront dorénavant plus obligatoirement soumis à ratification des parlements nationaux. Cette proposition de résolution européenne me semble équilibré dans la mesure où elle prend en considération différents aspects sensibles et différents points de vue en matière de commerce international et d'accord de libre-échange, elle reflète à cet égard la sagesse de cette assemblée et je veux comme d'autres l'ont fait avant moi, saluer le travail remarquable de nos collègues rapporteur Pascal Alizart et Didier Marie. Ce que je note dans ce texte, c'est tout d'abord une approche globale qui est donc plus strictement centré sur le commerce stricto sensu ainsi la nécessité de l'intégration des dispositions contraignantes dans leur volet développement durable environnemental et social me semble être à cet égard novatrice fondamental, ça constitue une avancée, cela est d'autant plus important que comme il a été rappelé par l'exposé des motifs, ce ne sont pas les barrières douanières qui pose le plus question mais bel et bien l'ensemble de facteurs non tarifaires qui existe encore à ce stade. Ensuite, le texte accorde également une place importante à la problématique des produits sensibles, d'autres l'ont dit avant moi, mais en tant que rapporteur spécial du budget de l'agriculture pour la commission des finances, je suis convaincu de l'intérêt d'une telle prise en compte qui est, disons-le nettement, absolument nécessaire, la filière bovine, mais également celle des sucres spéciaux qui concernent nos outre-mer ne peuvent pas être balayés d'un revers de main, et je suis particulièrement satisfait que notre assemblée le rappelle explicitement à la Commission européenne lors de ce mandat de négociation, c'est également s'être esprit que je suis sensible à l'évocation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dans cette perspective, même s'il ne saurait s'agir de l'Alpha et l'oméga des politiques publiques en la matière. Avant de conclure, je voudrais souligner un dernier élément de cette proposition qui nous est soumise, dans un contexte d'essor sans précédent du poids des multinationales dans l'édiction mondial des notes dans l'édiction mondial d'énormes, je crois que la mise en place d'un tribunal bilatéral chargé du règlement des différends entre les États et les acteurs privés appelée de ses voeux par le texte serait de nature, bien entendu, à garantir le droit des États à réguler une telle disposition permettrait de répondre aux inquiétudes légitimes qui ont pu se faire entendre, lors de l'examen du TPP puis du CETA nous allons je crois dans le bon sens, en conclusion, comme vous le constatez, je suis favorable à ce texte, qui nous donne les moyens de peser dans les négociations qui vont s'ouvrir. Ceci ne doit pas empêcher le débat, je sais que nous discuterons avec profit de différents amendements visant en particulier à préciser le degré de contrainte que nous entendons fixée aux négociateurs certains amendements ont d'ailleurs été adoptée en commission afin par exemple qu'une évaluation exemptée des effets économiques et sociaux des accords soit réalisés c'est une disposition tout à fait opportune, mes chers collègues. Nous ne sommes pas à côté du monde en ce sens, je ne peux que vous inviter à réserver une issue favorable à ce texte, qui nous permettra de peser sur la séquence des discussions qui va s'ouvrir, merci de votre attention. Merci, la parole est maintenant à Monsieur Daniel Gremillet. Monsieur le président, Monsieur le ministre madame la présidente de la commission des affaires économiques, Ce Jean Bizet, président d'ailleurs l'affaire européenne, je voudrais bien sûr saluer notre rapporteur Anne-Marie Bertrand. Je, président de la commission des affaires européennes effectivement à travers vous remercier les 2 rapporteurs, ainsi que notre rapporteur ou type des affaires économiques du travail qui a été réalisé et surtout du contexte dans lequel il a été réalisé, effectivement, nous nous sommes prononcés le 18 janvier. Et depuis le 18 janvier les choses se sont accélérées, effectivement, je me félicite comme tous ici, que pour la première fois, c'est une première effectivement le Parlement peut débattre. Peut apporter toute la richesse des enjeux à travers ces négociations pour que la France puisse effectivement l'exprimer que l'Europe puisse effectivement s'en emparer, mais il y a en complet décalage entre ce qui s'est passé le 18 le le document sur lequel on s'est prononcé et les événements. 1er décalage c'est effectivement l'Europe qui se retire de plus en plus surtout les filets de sécurité. 2ème décalage, c'est le projet de texte suisse, suite aux états généraux qui fait apparaître de nouvelles contraintes de production en France 3ème décalage plus récent, c'est l'annonce au niveau de l'Union européenne effectivement d'une crainte et pour l'instant d'une non-position d'un non-positionnement clair de la France sur le budget de la future politique agricole commune, puisque il y a des scénarios qui vont jusqu'à une baisse très importante, au-delà des 15 et parallèlement à cela, en termes d'accord, nous avons 2 pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui effectivement affichent leur ambition. L'Australie affiche une ambition très libéral mais l'ambition aussi qui accompagne de manière significative à travers cette politique libérale, mais qui prend en charge, puisqu'à ne un accroissement de plus de 14 pourcent de soutien sur les contraintes environnementales que le pays peut émettre pour pour accompagner son agriculture la Nouvelle-Zélande qui annonce clairement une ambition pour le 2025 d'un accroissement de plus de 55 pourcent de l'exportation sur les produits laitiers. On voit bien effectivement et président la évoquée tout-à-l'heure Anne-Marie Bertrand aussi qu'on ne peut pas de ces négociations sans auditionner le contexte international, il y a les accords du 7 a eu des accords des discussions du maire et effectivement sud de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, notamment pour la filière bovine et la filière ovine en particulier, a un autre point je voudrais livrer dans le débat par rapport à ce décalage c'est effectivement les coûts de production, et c'est là qu'on voit effectivement notre responsabilité : responsabilité nationale en France et responsabilité européenne si je prends sur ce secteur de certains secteurs de production pour l'Australie, on a des coûts de production qui sont inférieurs à 70 pourcent de ce qu'on peut trouver au niveau de la France, alors je souhaiterais, Monsieur le ministre, qu'on trouve une cohérence entre le discours du président de la République à Rungis et le discours du président de la République à la Sorbonne, d'un côté, au niveau de l'affirmation de l'ambition européenne et de l'autre, effectivement d'une d'un affichage d'une politique française, nous sommes en totale contradiction avec les accords de libre-échange qui sont actuellement débattus, on ne peut pas, d'une part demander toujours plus de normes pour nos produits et ouvrir plus largement notre pays a des aliments qui ne reste respecte par les contraintes que nous nous imposons je souhaiterais à travers cette intervention dire tout simplement que la France et l'Europe doivent affirmer leur ambition, comme le font dans ces discussions, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, effectivement, il y a, pas question de se renfermer sur nous-mêmes le travail qui a été réalisé par les la commission des affaires économiques, notamment, et des affaires européennes et je reprends président Bizet complètement votre propos et doit s'inscrire dans la transparence, l'équilibre, la réciprocité et d'exigence au niveau normative et là il y a nécessité de respecter nos choix on ne peut pas d'un côté, avoir ses exigences normatives toujours supérieur supérieur qui ne respectent pas ce qu'attend le citoyen qui exigeaient au quotidien par les paysans qui effectivement nous mettent en situation de distorsion, alors effectivement, aujourd'hui, c'est une première Parlement associer au débat, a eu, à un an des élections européennes, ça peut avoir un sens pour redonner effectivement cette envie et ce partage de l'ambition européenne de cette construction européenne qu'il faut, il faut absolument réussir mais Monsieur mini c'est aussi un défi puisque, à travers l'expression du Parlement, il appartient maintenant à la France, effectivement, d'être clair, d'afficher ses ambitions européennes d'afficher sur les ambitions agricoles et faire effectivement qu'il y a une cohérence entre l'envie et la capacité à être supporté sur l'ensemble de nos territoires.

Indonésie. J'ai donc Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos 3 commissions compétentes ont adopté la proposition de résolution européenne relative aux directives de négociation en vue d'accords de libre-échange entre l'Union européenne d'une part, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'autre part à travers cette résolution, le sénat demande à faire valoir son point de vue le plus en amont aussi ses ses mains exercent une vigilance constante tout au long de négociations à venir, il va, il va aussi aux conditions de mise en oeuvre des accords déjà conclus et ceux qui le seront et ils sont nombreux, l'accord le plus emblématique, celui signé avec le Canada, communément appelé c'est-à-, il est entré en vigueur à titre provisoire le 21 septembre dernier d'autres accords ont été signés orange sont en cours de discussion avec Singapour, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie, le Mexique, Merck Voilà la frénésie de l'Union européenne a signé des accords commerciaux tout azimut, le président de la République française a demandé à ses homologues, un débat sur la stratégie commerciale de l'Union, et cela dans l'optique d'une Europe qui protège enfin des Européens pour y arriver, le président Macron veut freiner la signature de ce nouveaux accords de libre-échange et surtout mieux armé l'Europe contre le dumping social avec cette proposition, et quelques autres, notre président, il faut le reconnaître, n'a rencontré qu'un succès d'estime et pourtant le président Macron ne demandent qu'une politique commerciale faute sur l'équité et la réciprocité, si le président de la République tempérer la frénésie libre-échangiste de l'Union européenne, ce qu'il a des raisons, tout d'abord, il y a le problème de la forme, on se souvient que l'accord avec les États-Unis, communément appelé taffetas a été négocié dans le plus grand secret, en conséquence, il a suscité méfiance et défiance. Pour les accords à venir avec l'Australie et Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne, volonté de transparence nouvelle sauf qu'avec l'aide de bienvenue de la Cour de justice de l'Union européenne, les parlements nationaux n'auront plus approuver ces accords par prendra la précaution de ne pas soumettre des investissements Directs et les cours d'arbitrage avec une approbation réservée au seul Parlement européen, un Parlement national ne pourra donc plus bloquer la ratification d'un accord commercial dans ce nouveau format. Soit dit en passant, ce n'est pas très malin d'écarter les représentations nationales en pleine ratification du CETA, comme vient de le faire, le Parlement européen par l'adoption, le 26 octobre dernier d'une résolution qui va dans ce sens et si la commission des parlements européens veulent écarter les parlements nationaux de la ratification des traités, c'est parce qu'il y a de sérieux problèmes de fond, à commencer par la ville de contestation dans les traités commerciaux font l'objet de la part d'ONG, d'organisations syndicales et de représentants politiques et les accuse de négliger les normes sociales, la santé et l'environnement. Le CETA concentre sur lui toutes les critiques et compris les critiques sévères de la commission d'experts indépendants mis en place par le président Macron cet accord, disent ces experts est en totale contradiction avec les ambitions affichées par la France pour la protection du climat comme le défunt taffetas le CETA les accords en cours de discussion, non pas pour objectif de supprimer les petites barrières douanières existantes mais liquider les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes des pays d'Europe qui traduisent notre histoire économique nos rapports sociaux notre conception de la protection du consommateur, tout cela pour le plus grand bénéfice des multinationales de l'agroalimentaire et de l'industrie, la qui depuis des années, des accords de libre-échange ça multilatéraux, bilatéraux ont fait à ce jour le bonheur de la Chine et des multinationales, mais certainement pas le bonheur, ni de la classe moyenne européenne née des agriculteurs sans cesse sommée de s'adapter, en particulier les éleveurs certes l'Union européenne commence enfin à se protéger contre la Chine, tout cela donne tout de même l'impression que les multinationales arrivent progressivement imposer un nouvel ordre mondial dans lequel les états se réduit à l'impuissance et des citoyens réduire de consommateurs en conclusion : il faut qu'une majorité des parlements nationaux veillent à ce que l'Union européenne de pas en matière de libre-échange, l'erreur déjà commise indexe n'élargissement vers l'Est, c'est-à-dire se précipiter d'abord et réfléchir ensuite la résolution européenne, approuvée par notre commission démontre la lucidité de notre assemblée en la matière, je pense donc rapporter la résolution en l'état, éventuellement enrichie d'amendements qui vont dans son sens, je vous remercie de votre attention.

merci Monsieur le président, mes quelques remarques effectivement puisque c'est un débat est donc l'intérêt qu'on puisse interagir, donc j'ai bien entendu le défilé, prise de position forte des uns et des autres, je constate que, il y a quand même une relatif consensus qui s'est établi sur le texte, qui était présenté, et c'est vrai que c'est un texte, je trouve, voilà qui qui est équilibré, qui elle mérite de pouvoir montrer au niveau d'ailleurs européen hé bien une assez forte convergence de vue entre le gouvernement et le Parlement

le summum de nouvelle génération, et au contraire nous nous nous nous poussons pour avoir une nouvelle nouvelle génération si je puis me permettre, qui prennent en compte des enjeux à la fois justement environnementaux de droit social, etc, de telle sorte que effectivement notre ambition soit soit plus forte s'agissant des sujets de traçabilité, il est clair que nous souhaitons et nous sommes intransigeants sur les questions d'auditeurs, par exemple, il y a encore quelques semaines, a été dépêché une mission d'audit sanitaire aux sourds parce qu'on a tous en tête quand même ce qui s'est passé il y a quelques mois, quelques années et qu'il est hors de question effectivement de transiger là-dessus et donc de ce point de vue-là, le président de la République guère dans ce sur la Sorbonne appelaient à des outils renforcée en matière d'inspection d'audits etc. Vous évoquiez également le lait le sur le Japon, c'est un un, un élu qui va nous permettre de marquer des points pour un certain nombre de filières très clairement, donc je crois qu'il voit là, ne soyons pas en en défensif et voilà les puissances de l'argent, écoutez moi je crois qu'il y a aussi beaucoup de voilà de producteurs de filières qui ne sont pas forcément que des grands groupes qui puisse bien trouver des débouchés grâce à ces accords, et d'ailleurs tout danger c'est aussi après, il faut que ces accords sont conclus de faire en sorte que véritablement toutes les entreprises sur notre territoire, se rendent compte, hé bien des débouchés qui s'offre et donc là à chaque fois, je, je le dis haut aux chambres de commerce, je le dis, hé bien, à toutes les instances qui représente le monde entreprenarial il y a ce besoin de de faire savoir de d'expliquer, de, de, de montrer ses nouveaux débouchés, faute de quoi, ce sont d'autres qui vont s'en emparer, au sein de l'Union européenne, vous étiez plusieurs à évoquer naturellement le le secteur agricole, Pierre Louÿs Cyril pelle va en particulier et donc de ce point de vue là je veux dire que la France n'a pas à rougir, on a notre agriculture et l'industrie agroalimentaire au sens général naturellement et très à l'offensive au niveau international, je vous donne les les chiffre consolidé pour l'agroalimentaire en 2017 hein, augmentation des exports à plus de plus 6 pourcent avec un excédent à 6,2 milliards d'euros et sur les produits agricoles bruts, si on est en léger déficit en 2017 c'est essentiellement dû aussi à une récolte 2016, vous savez qui a été compliqué et très mauvaise à cause des intempéries notamment et que donc on on a 6 n'ont pas à rougir et et et de boues débouchés que serait d'ailleurs notre agriculture sans un certain nombre de débouchés à l'international, enfin moi j'ai en tête de l'export d'un certain nombre d'animaux de l'Yonne en Iran ou ailleurs, enfin bref, j'ai sur tout le territoire, j'imagine qu'on a des des cas très concrets et de ce point de vue là je vais rencontrer Christiane Lambert il y a 15 jours et et pour lui dire combien moi je souhaitais oeuvrer et je le fais au quotidien pour toutes ces filières au mois de décembre, c'était un embargo sur la volaille française donc j'obtenais la levée en Irak, dont 200 millions d'euros de marchés qui s'ouvrent à nouveau et donc je souhaite que ce travail, on le fasse avec toutes les les filières qui ont des groupes export et qu'on puisse se coordonner le gouvernement ces filières

L'Europe qui protège un État si a également été évoqué par plusieurs d'entre vous, Colette Mélot notamment et et André Gattolin, qui évoquait l'idée de de ne pas avoir de naïveté et et je peux vous dire que la la France est justement également à Bruxelles très sonore, très vocale pour hé bien demandez par exemple que les investissements étrangers puissent faire l'objet, et bien d'un d'une d'une d'un examen très attentif, il y a en ce moment des discussions d'ailleurs qui sont conduites dans lesquels on a réussi à emmener nos amis allemands, et puis il y a aussi cette idée que toute application mauvaise application des accords de libre- échange si on détecte des problèmes des anomalies puissent faire l'objet effectivement de de sanctions, l'objet de de mesures fortes et et de ce point de vue-là, on met l'accent aussi sûre, hé bien l'idée de de créer un un procureur commercial européen, ce qui, en bon français donneraient un chiffre renforcement de sa c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment va suivre au quotidien, alors il y a la négociation c'est un mais après les négociations, hé bien tout ça, ça doit se ça doit être suivie comme le lait sur le feu et il s'agit d'être intransigeant dès lors que on verrait que des dispositions ne sont pas appliquées ou mal appliquée et donc je crois qu'on a, on n'a pas une vision Angélique des choses mais bien une vision réaliste et je crois qu'effectivement si on est lucide : le vaste monde est un vaste théâtre des opérations, voilà comme on parle des opérations militaires, il y a, il y a peut-être des opérations économiques et que c'est bien de ce point de vue-là, la France doit se battre armes égales, donc il est hors de question de se désarmer, au contraire, on est plutôt dans logique de de réarmement était évoqué également les dispositifs liés effectivement à la au règlement des différends en matière d'investissement alors vous le savez la formule qui a été trouvé dans le CETA, est une formule qui est meilleure que l'ancienne SDS qui avait donné lieu à des débats dans cet hémicycle, d'ailleurs, mais pour nous, le stade ultime, c'est véritablement une cour permanente internationale qui permettrait d'avoir donc une instance qui ne soit pas juste une instance d'arbitrage mais vraiment qu'une instance pérenne

aux ambitions préserver donc c'est pas au rabais, loin de là : Stéphane Travert là réaffirmer un budget for pour la future PAC donc on on rentre pas dans la négociation en baissant pavillon, loin de là et puis s'agissant des là aussi, voilà je je renvoie tout ce travail qui va être fait avec avec les filières et et nous avons bon espoir d'être là, toujours à l'offensive, j'ai pas de beaucoup plus long, monsieur le président, parce que je crois que nous avons une douzaine d'amendements examinés et qu'il est déjà 23 de résolution européenne alors sur la résolution, j'ai 3 amendements en discussion commune le 12 rectifier, monsieur

Monsieur le président, Monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement reprend le point de vue du comité européen des régions que je cite : changer les règles du commerce international est un préalable indispensable pour relever les défis de l'agriculture, de l'alimentation et du climat le comité européen des régions demandent à l'Union européenne de peser de tout son poids de premières exportateurs et importateurs de denrées alimentaires pour modifier les règles du commerce international agricoles l'OMC 94 dans le sens de relations commerciales plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus durable la crise l'agriculture connaître un certain nombre de crises structurelles, notamment concernant le lait, la viande bovine, ou encore les sucres spéciaux dans les régions ultramarines l'alinéa 19 ne tire pas toutes les conclusions qui s'imposent concernant les accords de libre-échange en effet, il convient d'exclure toutes les denrées alimentaires, des accords internationaux de libre-échange et non seulement demandé aux négociateurs dit porter une attention particulière comme la rédaction actuelle demande mais, chers collègues, à terme, nous devons arriver à créer une gouvernance mondiale de l'alimentation, il est intolérable délaissé les denrées alimentaires essentiels à la survie des populations aux mains du seul marché libéral puissant, le droit à l'alimentation est un droit humain fondamental : la souveraineté alimentaire des territoires doit en être une garante, je vous remercie. Le 10 ce rectifier c'est un amendement de repli qui ne concerne que les denrées qui sont dans le texte. Merci toujours donc en discussion commune le 3ème Monsieur Merci monsieur le président. Bon, comme vient de le préciser notre Couet collègue Joël Labbé, nous souhaitons simplement que les produits sensibles soient exclus des négociations, tous notre agriculture, notre agriculture, pardon, sera la grande perdante de ces accords de libre-échange contenu de la différence dans le modèle d'exploitation, la filière viande bovine risquerait d'être ravagée en Europe en cas d'ouverture des marchés, cela est précisé dans le rapport, cela a été même soulevé par la commission agriculture du parlement européen qui a elle aussi demandé une exclusion claire des filières les plus sensibles de ces négociations, à commencer par les viandes bovines et ovines, les produits laitiers et les sucres spéciaux les parlementaires européennes considère aussi qu'une plus grande ouverture du marché dans ce secteur pourrait avoir des conséquences des Sastre pour les producteurs européens, il met en garde contre le risque d'un fort déséquilibre de ces accords dans le secteur agricole au détriment de l'Union européenne, comme cela est rappelé dans de nombreux rapports l'agriculture européenne est clairement dans une position défensive par rapport au produit Néozélandais et Australiens notamment des produits d'origine animale, en particulier au regard des coûts de production qui sont parmi les plus faibles au monde est lié à des pratiques extensive de plus, vu la taille des marchés de ces pays, l'intérêt offensif or OPL à des produits de niche et dépendent de la levée de barrières non tarifaires cela, nous sommes d'autant plus important qu'aucune évaluation n'a été faite des impacts des différents accords de libre-échange déjà signé sur notre agriculture, c'est donc le sens de notre amendement. Merci donc sur ces amendements, l'avis de la commission Madame Bertrand. Exclure a priori tous les produits agricoles sur cela revient à mettre une terme aux négociations commerciales avant même leur début, c'est une demande qui n'a aucune chance d'être acceptée ni par la Commission européenne, ni par les autres États-membres par ailleurs l'exclusion complète et les produits agricoles et contraire aux intérêts même du monde agricole français et européen. La France a par exemple des intérêts offensifs, or dans le domaine des veines, fait de la reconnaissance et des indications géographiques un objectif essentiel il faut bien entendu être très vigilants sur l'avenir des filières sensible mais il ne faut pas considérer l'agriculture française uniquement à travers le prisme de cette filière, nous avons intérêt à promouvoir les exportations agricoles et alimentaires, car la France a un gros potentiel dans ce domaine, concernant le cas précis des filières agricoles les plus fragiles, la proposition de résultats de résolution offre une réduction une rédaction beaucoup plus équilibrée et protectrice des intérêts français, que ce que proposent ces hommes dans la commission demande soit le retrait soit un avis défavorable. Donc vie défavorable sur les 3 amendements, Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Même avis je ne saurais mieux dire. Même avis. Donc je reviens donc au vote, donc il y a des explications de vote ou des retraits par rapport aux demandes. Monsieur l'abbé. Monsieur le Président Monsieur chacun avec le plus le 1er rang amendement aller très loin, d'une façon extrêmement volontariste, c'est un amendement d'appel je le retire celui-là mais je maintiens le second. Donc il nous reste 2 amendements au vote pas d'autres explications de vote, donc le 10 rectifier qui est favorable. Qui est contre. Qui s'abstient. Tout le monde n'a pas dû lever la main, un moment ou un autre, mais c'est pas grave. Il n'est pas l'adopter.

Comme nous l'avions déjà mentionné, dans notre proposition de résolution sur les conséquences du traité transatlantique pour l'agriculture et l'aménagement du territoire, l'agriculture est un secteur économique essentiel pour notre pays, depuis plusieurs années, connaît des difficultés croissantes et récurrente différentes filières en traversé des crises graves autrefois 2ème exportateur mondial derrière les États-Unis, notre pays est passée au 5ème rang, devancée par l'Allemagne, les Pays-Bas et maintenant le Brésil aujourd'hui la filière de l'élevage se trouve dans une situation critique, près de 10 pourcent des exportations étant au bord du dépôt de bilan et la filière les confrontés aux conséquences de la disparation des quotas d'une façon plus générale, l'agriculture n'échappe pas au désastre de mondialisation des échanges, de plus, l'accord de libre-échange avec le Canada prévoit déjà son lot de 50000 tonnes de viande de boeuf importé sans droits de douanes au profit de la Coupe du maintenant ce sont des quotas supplémentaires que la Commission européenne s'apprête à accorder à l'Australie, ainsi qu'au Mercosur, sans se soucier des conséquences pour nos éleveurs, l'emploi et la vie rurale, cette situation est d'autant plus inquiétante que la la gris culture est déterminante pour la cohésion territoriale de la France dans les zones rurales fragiles les difficultés des espaces passion menace la pérennité de l'activité économique qui leur sont liés comme les abattoirs, les services vétérinaires, les entreprises de transformation des produits mais aussi celle des services de proximité tels que les écoles, la présence postale ou les petits commerces, c'est donc le devenir de nombreuses communes rurales qui est un jeu, de même que la préservation de l'équilibre des paysages et des territoires, avec le risque d'extension d'Éric défriche ou défaut et c'est pour ça, c'est pourquoi nous souhaitons qu'une attention particulière soit portée sur la ruralité. Merci l'avis de la commission Bertrand. car des accords commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne mettent pas en danger de la sauvegarde de la société rurale de son économie et de son identité, le laisser penser, comme marin exagéré, il y a même de fortes chances que certaines filières agricoles françaises tirent profit d'telle accords notamment la filière vinicole, ce qui est vrai en revanche c'est que la négociation de ces accords, M. Picot comme prête une attention particulière à certaines filières agricoles fragile et qu'en mettant en place des mesures de protection adaptée à ces filières sensible, c'est ce que fait cette proposition de résolution européenne. Même avis. Et s'il y a des explications de vote, pas d'explication de vote donc je mets l'amendement numéro 6 aux voix qui est pour. Qui est contre. Abstention donc l'amendement n'est pas adopté. Le 7 monsieur qui toujours. Merci monsieur le Président, je repars de la chance, comme ça été précisées en commission, vous le comprendrez, c'est un amendement d'appel mais je crois que il il a le mérite d'avoir le débat. la République le de la République, Emmanuel Macron ça à une transformation de la politique commerciale européenne pour une Europe qui protège et la Commission continue de dégoût aussi une série d'accords de libre-échange qui mettent en danger les droits sociaux et la protection des consommateurs, l'environnement et nos principes démocratiques principes démocratiques, car même s'il y a un effort de transparence, celui-ci reste limité, selon les termes du rapport de la commission des affaires économiques de plus pour contourner la jurisprudence de la Cour de justice sur les accords mixtes et donc la compétence des États-membres, la Commission européenne a décidé de samedi, les négociations afin d'asseoir sa compétence est-ce plus veut comme nous l'avons déjà mentionné dans notre intervention General c'est pourquoi, par exemple, règlement des différends ne fait pas partie du mandat de négociation, il en est lui-même de du chapitre sur les investissements, elle pourra dès lors faire adopter ces accords de libre- échange sans consultation des États-membres ainsi ce seront des traités négociés dans des conditions de très éloignée des principes de traces par un c'est de contrôle démocratique qui vont encore une fois déterminée en grande partie l'avenir de notre agriculture et de l'aménagement du territoire, dans les pays membres, la politique agricole française a jusqu'à présent cherché à concilier la modernisation avec les objectifs de maintien de l'exploitation familiale de qualité et de diversité de la production d'aménagement équilibré du territoire et d'entretien du paysage, les négociations de cours pourrait conduire à une profonde remise en cause de notre schéma, l'école et à des changements économiques profonds, c'est certaines gares ne choix de société, il n'est pas acceptable, selon nous, que ce choix soit aussi lourd ne fassent pas l'objet d'un débat que démocratique, c'est donc le sens de notre amendement. Bien sûr, cet amendement numéro 7 madame Bertrand l'avis de la commission. Donc cet amendement se heurte à un obstacle juridique de taille la Cour de justice de l'Union européenne a rendu le 16 mai 2008 17 E n'important d'avis qui permet de préciser à quelles conditions un accord commercial et mixtes ou non. Très clairement, ce compte tenu de sa et clarification par la Cour de justice de la portée des traités européens en matière de politique commerciale qui a pour effet d'exclure l'approbation finale des accords par les États-membres et deviennent plus que jamais et c'est ainsi de peser sur les accords en amende de leurs conclusions et je vous le demande, Monsieur le Ministre, il n'y a plus de possibilité de véto national au stade de la ratification donc retrait sinon avis défavorable. avait du gouvernement. Même avis pour le gouvernement, donc je vais mettre cet amendement numéro 7 au revoir monsieur Guy, explications de vote. On est là pour débattre, même si l'État, je sais bien mais c'est pas moi qui choisi l'horaire, je vais pas être plus long mais ça mérite qu'on a un débat profond. En tant que parlementaire, est que nous pensons que nous n'avons pas notre mot à dire sur ce traité de libre-échange, je note la progression, il y a maintenant une clarté sur le mandat qui est donnée, c'est une bonne chose, nous l'avons exigé jusqu'à présent, ça se négocier au 3ème sous-sol de la Commission européenne et nous n'avions rien à dire, mais une fois que nous avons la mandat clair est-ce que à la fin il m'apparaît. je pense réelle mais on peut avoir le débat, je, je, si je suis minoritaire, je me plierai mais est-ce que nous pensons comme tant que parlementaires, nous n'avons pas notre mot à dire sur la fin des logos Et quand on a ce débat-là, certains nombres d'entre nous disent oui, alors j'entends les aspects juridiques, je les connais comme vous, mais je crois que si le jeu, le juridique n'est pas bon, il faut que nous ayons ensemble. Une action pour changer cela. Nous allons pas à chaque fois, nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon que on va se replier derrière juridique si ce n'est pas bon alors, agissant pour le faire, il est normal que certains nombre de parlementaires, mais des 27 États-membres et leur mot à dire et donc c'est ce débat-là que je veux qu'il soit public avec cet amendement, donc je vais pas le soumettre au vote, je vais le retirer parce que j'entends l'argument juridique, mais je pense qu'il faut que nous ayons un débat assez profond, alors j'entends, il est minuit, mais je pense que c'est un débat qui va traverser les prochaines semaines et les prochains mois et donc, j'espère, Monsieur le Ministre, à cette occasion je pour entendre votre voix sur cette question là. Donc là, Monsieur Bizet voulait intervenir. Oui, monsieur le président Monsieur Miss mon cher collègue, je ne voudrais absolument pas allonger les débats, je ne prendrai qu'une fois la parole sur l'ensemble des amendements mais vous avez eu je dirais le la pertinence de rappeler en toute dernière intervention que juridiquement, vous aviez tort parce que ça relève du traité de Lisbonne et, précisément, si vous voulez, sachez que le Parlement européen et lui seul sera appelée à se prononcer, c'est quand même assez démocratique et le Conseil de l'Union, là aussi c'est c'est démocratique, ceci étant, le Sénat est pratiquement la 1ère chambre, si vous voulez avoir très en amont, avant d'avoir, je dirais, au travers de la directive une définition du mandat clair de négociations, un débat et moi j'avais toujours souhaité, plus on aura des débats en amont, plus on aura des débats pendant les négociations, plus ce sera facile d'expliciter sur le terrain et je ne voudrais pas qu'on se retrouve, si vous voulez dans la même configuration dans la même posture que la Wallonie, où on a eu une très mauvaise image pour lait pour l'Europe pour pour les négociations de 2 mots, également par rapport aux amendements précédent qui qui qui n'ont pas été retenu quand vous avez parlé de la société rurale de soi ne peut nommer de son identité faut rappeler que 30 pourcent des emplois dans l'agro-alimentaire concerne précisément les politiques de l'exportation comme vous avez appelé à l'identité des zones rurales, il faut savoir que la protection des indications géographiques, c'est précisément la protection et la vitalité de de ces zones rurales, on pourrait continuer et juste un mot sur la filière viande rouge parce que

à se réformer, c'est vrai qu'elle risque d'être fragilisée mais ce qu'il est normal que 2 pourcent de la production bovine française soit soit contractualiser, c'est quand même un peu un peu de la viande qui passent en ira chef et de la viande d'importation que 45 pourcent de la viande transformée en France va en steak haché il faut réformer cette filière, le fonds d'adaptation de la mondialisation fait aussi pour ça, il ne l'est pas, aujourd'hui, il faudrait qu'il le soit et on pourrait continuer les, les, les explications si vous voulez, mais quand monsieur le ministre a dit tout à l'heure aussi que, aujourd'hui, si vous voulez, la balance commerciale au niveau de la grille agroalimentaire en 2017 était de l'ordre de 6,2 milliards je voudrais lui rappeler qu'il y a 2 ou 3 ans, elle était à 8 milliards et quelques, donc faisons attention de ne pas fragiliser notre tissu agroalimentaire au détriment de pays qui sont extrêmement importateur sans les mêmes signes de qualité sans les mêmes si, si vous voulez, je dirais, de valeurs, de nos produits, à savoir l'Allemagne et les Pays-Bas.

et s'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé donc l'amendement suivant, c'est le 11 rectifier, monsieur l'abbé.

c'est une question de démocratie, monsieur le Président, Bizet, quand je vous entends parler, je me dis : on ne parle pas le même langage, on n'est pas de la même planète je suis désolé, je ne défends pas les mêmes valeurs que vous vous êtes brillant dans vos, manière de dire les choses, mais derrière ça, il y a des rats et des réalités, il y a des réalités de terrain, il y a des réalités humaines, il y a des règles, des réalités de droits humains, alors je n'irai pas plus loin, je retirerais même mon amendement, mais il reviendra un jour ou l'autre bien sûr.

Oui, Monsieur le Président, cet amendement a pour objet de remplacer l'alinéa 27, telle que proposée dans la PPR heureuse, nous l'avons déjà défendu à 2 reprises en commission et il vient d'obtenir un avis favorable ce matin lors de notre réunion il reprend mot pour mot la position des autorités françaises actuelles portant spécifiquement sur la perspective de l'ouverture des négociations commerciales de l'Union européenne avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, rappelons ici que notre abonnement propose, il préconise de systématiser au niveau européen, les évaluations en amont des projets de négociations et que celle-ci puisse tenir compte des négociations en cours ou récemment conclu afin d'éviter l'impact cumulé des accords commerciaux sur les secteurs les plus sensibles. Avec la multiplicité des accords en cours de négociation, il est essentiel aujourd'hui d'aller au-delà du simple rapport de la Commission européenne, faisant état de négociations en cours, comme celui qui a été publié le 9 novembre 2017 et de la publication d'études d'impact accord par accord. contexte, dans ce contexte opportun de disposer au niveau européen, d'un document qui fasse l'état des secteurs et des produits par filière et par États-membres en amont des négociations permettrait de disposer d'une vision globale sur les marges de négociation, de renforcer nos positions de négociation, de mieux prendre en compte les fragilités spécifiques à certains secteurs, à la fois au niveau européen et par États-membres et d'éviter ainsi expose les risques de déstabilisation durable de filière entière qui seraient touchés concomitamment par plusieurs accords, les autorités françaises dans leur note de position de janvier 2010 villes précise ainsi qu'il convient désormais de prendre aujourd'hui, je cite, des initiatives visant à améliorer la méthode de négociation pour créer la confiance nécessaire au 1er rang desquelles figure la nécessité en amont des négociations de ce travail d'évaluation, je vous demande donc de soutenir cet amendement. Oui, donc l'avis de la commission Madame Bertrand. L'avis de la commission est favorable. L'avis du gouvernement amendements ayant été puisées à bonnes sources, le gouvernement est favorable. Très bien, donc l'amendement numéro 4 que je vais mettre aux voix, s'il n'y a pas de d'explications de vote avec 2 avis favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Oui, effectivement, c'est un amendement qu'on a écrit avec Laurent du plomb et Alain Châtillon républicain Union centriste, je comprends bien qu'il dérange un peu. Mais l'Europe a construit des normes de production et des qualités de produits européens, il faut que les produits importés correspondent aux mêmes normes c'est l'objet de l'amendement, donc on demande aux négociateurs que tout nouvel accord de libre-échange soit établi sur l'exigence de mise en oeuvre de normes de production comparables, a fait l'de l'Union européenne concernant les produits destinés aux consommateurs de l'espace communautaire cela tant au niveau des normes sanitaires, phytosanitaires environnementale facial qu'au niveau des normes relatives au bien être animal et aux prescriptions de la dénomination de vente.

Et effectivement Monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est un sujet qui est relativement important par rapport au débat qu'on a et la rupture qu'il peut y avoir de compréhension entre des discussions sur les accords qu'on peut passer entre l'Union européenne et un certain nombre de pays aujourd'hui, nous venons de terminer Madame la Présidente Commission économique des affaires économiques, un long parcours d'auditions sur les affaires de la salmonelle et on voit bien les exigences qu'il y a aujourd'hui au niveau de la société et et du consommateur, et il est essentiel, effectivement, pour que dans le cas de discussion équilibré qui a un respect de ses attentes à la fois du des citoyens des consommateurs par rapport aux produits importés, c'est vraiment essentiel et c'est aussi l'notions d'équilibre puisque dans ces accords, je prends des exemples sur la Nouvelle-Zélande, notamment il y a dès précautions sanitaires en matière d'importation de produits agroalimentaires en Nouvelle-Zélande qu'il faut aussi respecter, donc il y a des choix qui appartiennent à ces espaces d'échange à l'Union européenne, qui est une belle chance pour l'agriculture, effectivement, il y a d'énormes et c'est dans ce cadre-là qu'on veut nous considérons que le mandat et le désengagement d'Union européenne doivent être réalisés, c'est vrai pour les agriculteurs européens, mais ça doit être vrai aussi pour qu'il a pas tromperie sur les produits qui seront importés en concurrence des productions européennes et j'en profite, même si c'est pas le sujet mais j'en profite que monsieur ministre et là c'est l'occasion aussi de rappeler que si on veut une Agropur françaises performantes, il y a vraiment intérêt à ce que la France ne sur transposition parce que la surface position d'énormes apporte des contraintes supplémentaires, je dis : on est à la veille de débats sur la suite des états généraux et on voit bien que la France va remettre encore une couche supplémentaire sur le bien être animal, donc des des conditions de contraintes de surcoût qui peuvent mettre en situation de plus grande fragilité encore notre gré économie agricole rural et, bien sûr, toute l'activité donc et respect pour à la fois l'exigence économique mais surtout l'exigence de compétitivité qui est supporté par les acteurs économiques que sont les à les agriculteurs notamment, mais c'est un peu dans d'autres domaines, être vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité. Merci monsieur monte, j'ai souhaité la parole. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Je voudrais évoquer ne un sujet qui n'a pas été abordé dans les réunions de de commissions et qu'à traiter le président disait lors de la session du Sénat 4 80 1999 2001, il s'était intéressé dans le cadre d'un RAM ports d'information au Codex Alimentarius. Quèsaco comme on dit chez moi. Je pense que certaines entre vous connaissent ce ce dispositif, la commission qui le fait vivre Codex Alimentarius cette ce dispositif s'inscrit comme un organe commun entre la FAO et l'Organisation mondiale de la sainteté et il édicte des normes qui touche toutes en particulier à l'alimentation et à la sécurité de l'alimentation, donc il a l'objectif de protection de la santé des consommateurs les ainsi s'assurer, entre autres, des pratiques loyales dans le cadre du commerce international, ma question s'adresse à Monsieur le le le ministre, les instances européennes, siège dans cette instance dans cette commission Kahn est-il de la question des de l'harmonisation des normes à l'échelle R national à ce sujet et il y a bien entendu un rapport Direct avec l'amendement qui viennent de nous être présentées le ministre pouvez nous donner quelques éléments là-dessus et peut-être aussi le président Bizet qui connaît parfaitement ce ce sujet ça pourrait nous éclairer et ça pourrait aussi constituer non pas pour pour le texte de de ce soir, mais pour nos travaux ultérieurs, une piste de travail peut-être intéressante et fructueuse. Merci donc, explications de vote Monsieur Merci Monsieur le Président, juste parce que ça méritait débat mais puisque vous l'avez évoqué, monsieur le président de la Commission européenne, traité de Lisbonne, tout ça, je suis au courant, j'ai vendu à l'époque du traité de Rome, qui en fait le copier/coller, que nous avons refusé à 55 pourcent des centaines d'exemplaires de l'Humanité dimanche, à l'époque pour bien que nous comprenions et donc il me semble un peu bizarre de dire nous avons le traité de Lisbonne et nous sommes contraints par cela et c'est absolument démocratique, je vous dis, je n'ai absolument pas la même vision que vous mais ça mériterait débat, j'aime bien sûr l'amendement, je vais le voter. Je crois qu'on va être nombreux à le faire, mais je le dis, c'est pas le même cheminement intellectuel et politique qui m'amène à le voter. Mais je, je pense qu'il est intéressant. Pourquoi, parce qu'il dit, on voit bien, moi je ne cohérence. Mais au sein bien qu'il y a des contradictions, y compris de personnes qui disent je dis pas que c'est les auteurs de l'amendement attention mais entre certains qui disent, laissant le faire le libre-échange, partout, on verra bien, tout va s'autoréguler ouvrons tout surtout aux capitaux pas aux être humains et y compris je suis pas pour qu'on ne caricature ma position, moi je suis pour découper rations pour les peuples. Je dis pas qu'il faut se replier sur lui-même. Ce repliés sur nous-mêmes et pas pas faire marcher avec d'autres, mais il faut des normes. Et je suis satisfait, enfin c'est un 1er pas cet amendement parce que y compris, je suis pas pour le moins disant social et environnemental. Je suis pour le mieux-disant social et environnemental, partout dans le monde, quand je parle de coopération entre les peuples et par exemple sur nos produits. tickets le viande ovine, etc, je suis pas pour que nous-mêmes nous profitions des systèmes de l'autre côté du monde qui pressuriser des agriculteurs et des agricultrices Les les coups bas, je suis pour que nous, et le viande tout ça et donc c'est à une première étape, je dis ça, je dis que, il faut que nous menions une comment appliquer un combat politique, je l'entends bien à l'échelle mondiale, mais pour que les normes. Pour nous, que nous souhaitons déjà homme roux au niveau européen. Nous les partout dans le monde, donc je le voterai voilà et j'espère que un certain nombre d'entre nous, je pense que nous aurons l'unanimité. Oui, explications de vote toujours monsieur Bourquin. Oui, monsieur le président Monsieur mini-ses chers collègues, je voterai aussi c'est un amendement d'amendements qui demande une réciprocité d'énormes entre l'Union européenne et les contractants des traités. Sinon comment nos entreprises à qui on met des normes beaucoup de noms. ça coûte cher. C'est aussi la productivité si à côté vient se vendre des produits. Qui n'auront pas les mêmes exigences dans les accords, s'ils ne prennent pas en compte cette dimension inévitablement peuvent coûter cher à l'industrie française, mais aussi à l'agriculture française, à quoi Servent ces traités ces traités ont une ambition, c'est les avantages du libre-échange, baisse des prix. Des biens et des services, augmentation de la croissance et tout cela, il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence beaucoup plus forte des produits et que ceux qui ne sont pas capables de supporter cette concurrence inévitablement s'arrêteront imaginez dans une filière comme le lait, ce qui peut se passer, imaginez dans les filières de la viande qui est la plus comment qui est la plus soucieuses de ce qui va arriver et, inévitablement, il peut y avoir aussi pour faire face à la concurrence, une volonté de faire baisser les acquis sociaux. Qu'est-ce qui a dit : je pense qu'il y a une fuite en avant de la Commission dans la signature des traités de libre-échange qu'est-ce qui a dit ça Emmanuel Macron. Emmanuel Macron il l'a dit, lorsqu'il a visité Rungis et au contraire, j'ai vu le lendemain la le président de la Commission européenne, qui a dit : mais non, il y aura le Japon alors à Singapour et et c'est pour ça que c'est un moment est important, une volonté, si ces traités se mettent en place, qu'il y a un équilibre entre les normes françaises et l'énorme avec lesquels on commerce sinon on charge la mule, comme on dit, on est en train de naître des repas handicap à l'économie française et à l'économie européenne et au bout, on aura beaucoup de perdants et pas de gagnant, ça doit être dans le mandat.

et souvent, la commission a été mise en cause sur ses exigences de réciprocité, on va pas comme ça aux États-Unis, on va pas comme ça au Japon. Et on doit avoir une volonté de de réciprocité. Merci monsieur l'abbé.

vers le haut la question des normes sanitaires et finaux et phytosanitaires, elles ne vont pas aller en diminuant, ce ne sont pas les résultats d'hier sur des prélèvements qui ont été faits sur les produits phyto-sanitaires sur des fruits et des légumes en France qui vont faire aller vers le bas, on doit être plus exigeant encore Daniel Grébille a évoqué la question du bien-être animal, il faut savoir que les questions de bien-être animal ne vont pas aller en diminuant non plus alors justement, cet amendement est drôlement intéressant parce que nos partenaires économiques auront lieu de s'aligner sur l'Europe et Kandziora Pierre plus ou encore souvent entraînés par la France. Eh bien, c'est l'ensemble de la de la population de la planète qui en bénéficiera.

moi je suis absolument en phase avec l'esprit entre guillemets de cet amendement, je le suis moins sur la rédaction, notamment sur la 2ème ligne parce que je pense que il y a un petit problème de cohérence et un petit problème également de langage communautaire, commentent les auteurs écrivent l'exigence de mise en oeuvre de normes de production comparables, ce serait plus communautaire et et et cohérent de mètres l'exigence de normes tout simplement comparables parce que si vous voulez c'est accords commerciaux de 3ème génération on a essentiellement pour but si vous voulez de maîtres-à terme en cohérence Les Les les barrières non tarifaires et la la rédaction n'est pas tout à fait je dirais communautaire voilà moi je, je le dis, bon, j'en fais pas un casus Belli, mais à mon avis, vous seriez plus entendu par la commission si je puis dire, en mettant simplement l'exigence de normes comparables, ça c'est le 1er point

c'est vrai que c'est une terminologie qu'on utilise plus beaucoup, c'est un tort, c'est un tort, parce que c'est véritablement une bible est une référence qui est partagé à la fois par l'Organisation mondiale du commerce et la FAO, la foi d'un agriculteur l'organiser ce sont des normes qui sont régulièrement mises je dirais à niveau puisque, en fonction de l'évolution des je dirais des acquis ou des connaissances scientifiques, elles sont régulièrement mises je dirais c'est vrai que on y reviendra sur ce type d'accord, si je puis dire, hein, pour la bonne raison, c'est que ça durera des années et plus on aura de débat ici au Parlement, plus on encadrera entre guillemets les éventuelles dérives de la commissaire, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, enfin en ce qui concerne les normes européennes, encore une fois, moi j'ai vidé de mon intervention préalable, ce qui serait souhaitable, c'est que, et c'est ça, c'est l'objectif également du président c'est que on peut peut-être être un petit peu perturbés par la volonté de l'Union européenne de multiplier les accords de libre-échange des accords bilatéraux pourquoi bilatéraux parce que, de façon le multilatéral est en panne, donc en objets d'en faire plusieurs, pendant que les États-Unis sont en période de je dirais de crispation et de protectionnisme, plus on pourra faire avancer les normes européennes, plus on a de chances que ces normes européennes deviennent les normes de référence mondiale, et je préfère les normes européennes aux normes chinois, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur le président merci donc je pose la question à l'auteur, représentant du moins de l'amendement monsieur lourd est-ce que vous acceptez cette modification. je propose effectivement un sous-amendement qui prend en compte et qui dit mise en oeuvre de normes comparables à celle de l'Union européenne, mais non pas voilà, nous l'acceptons mais mais il faut vraiment que Léo fonctionnaires fait que ce qui vont négocier comprennent que l'agriculture européenne est bâtie sur des exigences européennes sur des exigences de qualité sur des exigences de normes sur des exigences de consommateurs et qu'aujourd'hui les habitants de l'Europe sont en droit d'attendre et c'est à l'Europe de tirer vers le haut la qualité de sa production mondiale. Donc, c'est simplement une une une modification de de rédaction du texte, c'est pas en être un, un sous-amendement dans la mesure où le sens n'est pas n'est pas modifié simplement l'utilisation de mots, je pose quand même la question à la Commission et au gouvernement s'il n'est pas d'objections sur cette modification, très bien très bien monsieur le ministre est également favorable, ça va dans le sens de l'ensemble des intervenants, donc je suppose qu'il n'y a pas de nouvelles explications de vote compte tenu qu'on se dirige vers quelque chose. De relativement consensuel, donc l'amendement devient la demande mon rectifier Water et je le mets aux voix qui est pour. C'est contraint. Qui s'abstient donc l'amendement et est adopté. L'amendement suivant, donc ce qui est ce qu'il défend Monsieur nouveau, toujours le 1 rectifier terre. Eh bien là tout simplement les négociations, c'est du Business, et dans le Business, il faut des hommes d'affaires et on a l'impression que dans les négociations, les hommes d'affaires concernées ne sont pas au côté des négociateurs et on propose de demander aux négociateurs, compte tenu de la complexité des enjeux d'être accompagné lors des discussions désaccord de libre-échange 2 personnes dont l'expérience et la compétence font autorité dans les domaines concernant concernés par cet accord.

dans la vraie vie, je vois pas comment ça se passe, ce que je veux dire, c'est que les négociateurs, il vont pas venir avec les 27 MEDEF

comment dire, il consulte et moi je peux vous dire que les tous les secteurs concernés rencontrent très régulièrement les négociateurs, les services de la Commission pour faire valoir leur point de vue nous-mêmes au niveau national, on le fait, donc, en réalité, enfin je je comprends l'attention de l'abonnement, c'est que, c'est que les négociateurs soient pleinement éclairés mais mais dans la vraie vie,

des avis positif et favorable, essayons de le garder le plus pur possible et et et on comprend votre attention, mais je pense que voilà,

Que les négociateurs ne sont pas très dur avec les partis qui sont en face, et voilà, c'est fini. Monsieur monsieur

alors si on veut les introduire carrément dans les négociations, à quoi ça sert d'avoir des représentants et d'avoir des représentants élus et d'avoir aussi un corps qui s'appelle les diplomates et haut fonctionnaires, je pense que on peut dire, il peut y avoir des consultations peut poser tout ce qu'on veut mais ce n'est pas aux chefs d'entreprise de négocier, ils ont d'autres contrats négociés personnellement.

Donc la commission a émis un avis favorable, même si personnellement j'étais pas favorable, Très bien, donc avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement, il n'y a pas de d'explications de vote supplémentaire Monsieur Gay. Pour une fois je suis d'accord avec mon collègue d'en marche. C'est rare, mais des fois ça arrive. Il est minuit, bon c'est c'est c'est une question moi j'entends qu'on est des gens sérieux et je partage votre avis. Je suis pas d'accord politiquement. Mais on peut pas dire que les gens ne sont pas sérieux, ils vont négociations ils appliquent ce qu'on leur a demandé politiquement. Je suis. Il faut faire attention, bon, on a beaucoup de questions sur les lobbies.

y a personne dans l'expérience et la compétence font autorité dans les domaines concernés par ces accords. Les premiers noms qui vous sont venus à l'idée, c'est le MEDEF et les entreprises, mais vous savez, par exemple dans les Syndicate salariés il y a beaucoup de gens comme des choses à dire, et comme beaucoup de compétences équipe aussi pourrait aller au terme des négociations et pourrait dire beaucoup de choses, voilà, mais c'était juste un petit club. Merci, Monsieur le Ministre. En réponse à monsieur, il y a, lui dire que justement dans le comité de suivi de la politique commerciale, nous associons les syndicats et plusieurs représentants des syndicats sont présents.

Et je reviens à l'amendement 3 édifié bis Madame Mellow. Merci monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le Ministre, cet amendement a pour objet d'appeler la Commission européenne à prévoir des dispositions relatives aux services numériques, encourageant les flux de données transfrontière, tout en assurant le respect de la législation européenne en matière de protection des données et en prévoyant un droit des partis à réguler ce dernier point important face à la vision anglo- saxonne de libre circulation totale des données recueillies réduisant la capacité des États à réglementer un rapport de l'Inspection générale des finances de 2016 relatifs aux enjeux numériques des accords sur le commerce des services préconisé d'adopter cette précaution à l'avenir tout un encourageant la circulation des données entre les parties des accords dits d'adéquation Régis, par ailleurs, le transfert de données personnelles entre l'Union européenne et l'Australie, ainsi que la Nouvelle-Zélande.

Oui c'est un avis favorable à cet amendement, je crois, permettra justement de peser face à une vision un peu anglo-saxonne de la libre circulation totale des données, ce qu'on appelle le Free-flow of Data dans la langue de Molière,

les accords de libre-échange, nous l'avons même fois répété ne sont qu'une fuite en avant. Où il y aura de nombreux perdants, outre une énième déstabilisation des filières, le risque est celui de l'industrialisation des fermes, donc d'une augmentation importante du foncier agricole dans les zones concernées d'une concentration géographique par spécialisation et en définitif d'une désertification et d'une dégradation de nombreux territoires ruraux, l'agriculture et agroalimentaire ne doivent pas être les variables d'ajustement de la négociation de ces traités les accords de libre-échange ne peuvent être prétexte à nivellement par le bas au démantèlement ou allait faiblissent manque de toutes les normes qui limite les échanges même les normes sociales ou environnementales, c'est pourquoi nous pensons que tout accord doit être subordonné au maintien de où niveau de sécurité sanitaire pour les consommateurs et à la préservation du secteur de l'élevage en France que la France doit pouvoir soutenir une politique agricole ambitieuse sans risquer le couperet de l'interdiction des aides de l'État. Merci donc la vie de la Commission sur cet amendement Madame Bertrand sur le 9. Sur le 9 c'est un avis défavorable, parce qu'en fait il me semble que la plupart des points abordés dans cette abattent cancer la définition et l'évolution de la politique agricole commune, c'est un problème interne à l'Union européenne, le contenu de la PAC ne se défini pas dans le cadre de négociations commerciales avec des pays tiers, il ne faut pas se tromper de débat. Mais du gouvernement. Ne voulait pas finir ce débat sans apporter une réponse à l'un des amendements de Monsieur Guey façon détaillée. Et précise : voilà. Non mais donc ça sera l'avis défavorable, tout simplement parce que, s'agissant de de toute la dimension agricole, nous, nous pensons qu'il faut véritablement aller vers ce que la la la, commission d'ailleurs affirmé que l'amendement quel adoptée, qui est, cette enveloppe globale ce niveau maximum ce plafond de de concessions pour les les filières et puis après, ben ce plafond il est réparti entre les différentes négociations mais s'imposera l'Europe à faire ses propres arbitrages vis-à-vis de des eaux une tierce, avec lesquels elle négocie et donc il nous sommes que c'est la la voie la plus réaliste et puis intelligente qui qui mêle la prévisibilité dans le dans le système, s'agissant des normes de haute qualité, vous savez que justement le fait d'aller verser traité de nouvelle génération, même s'ils sont encore imparfaits et et qu'on conçoit les parfaire, c'est ce qui s'était dit, hein, c'est, c'est ce qui va nous permettre aussi de faire en sorte que nos normes soient peut-être plus universel que ce qu'elles ne sont et d'ailleurs, je vois bien avec le Canada sur les ça nous amène aussi à des poussées sur des sujets de bien être animal, ça, c'est aussi un levier pour faire en sorte que les mêmes évoluent dans leurs, dans donc un avis défavorable, maintenant voilà je je peux comprendre la cohérence de votre position au regard des amendements précédemment déposée mais le gouvernement également sa propre cohérence et donc ce soir ne se rencontrent pas tout à fait, mais en tous les cas, le débat a eu lieu, c'était tout à fait important.

parce que on peut s'inspirer aussi de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, je voudrais prolonger votre propos Monsieur Ministre parce que ça va dans un sens effectivement que d'autres pays peuvent s'inspirer des avancées significatives que peut faire l'Union européenne sur un certain nombre d'initiatives en au niveau des normes dès lors qu'elles sont réciproques, mais à l'inverse, sur des plans stratégiques, je prends la Nouvelle-Zélande qui vient ou les pouvoirs publics viennent de décider de financer sur 250000 hectares des plans d'irrigation pour améliorer la productivité sur ces territoires, la France pourrait s'en inspirer, avec des retenues nous, gestion de l'eau plus offensive qui permettrait effectivement d'avoir une meilleure compétitivité je, je le dis en passant, parce que c'était l'occasion certes dans les 2 sens monsieur milices, on peut aussi s'inspirer du volontarisme de certains pays, la France a cette chance, donc c'était dommage de ne pas le placer. Très bien, pas d'autres explications de vote n'était pas totalement une d'ailleurs, mais bon c'est le c'était en plein dans le sujet. Donc je mets au voile amendement numéro 9 avec avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Monsieur le Président. Cet amendement a pour objectif d'inviter le gouvernement à défendre, élaboration d'une stratégie commerciale commune consolidée qui intègre les exigences défendu dans cette proposition de résolution européenne l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mai 2017 sur l'accord, Union européenne, Singapour a conforté la compétence exclusive de la Commission sur la négociation de tous les volets des accords commerciaux, à l'exception du mécanisme d'arbitrage en matière d'investissement. Le groupe socialiste considère en conséquence que les États membres et la Commission doivent à nouveau arrêté en amont une nouvelle stratégie de politique commerciale reposant sur un corpus commun d'exigence et de principe valable pour tous les futurs accords commerciaux conclus par l'Union européenne. La France a d'ailleurs demandé au Conseil européen d'octobre 2017 que ce travail soit engagée en particulier en ce qui concerne les exigences de dispositions contraignantes en matière de développement durable le mécanisme arbitral nouvelle forme une pour les conflits États investisseurs, elle a également remis un an Pepper au Conseil, à l'Automne pour, je cite, de redéfinir la politique commerciale européenne dans l'intérêt de l'Union et des États membres et présente un certain nombre d'initiatives, notamment en en matière de méthodes de négociation qui rejoint les préoccupations et les exigences de cette PPR pourtant, pour l'heure, aucun débat formel n'a encore eu lieu au Conseil sur l'opportunité de consolider cette stratégie, ce que le gouvernement français a d'ailleurs regretté en janvier dernier, et donc il est du devoir du Parlement de peser de tout son poids pour que ce débat est lié au conseil. C'est le sens de notre amendement qui a recueilli un avis unanime de sagesse en commission et bien entendu, nous formons des voeux pour qu'il soit définitivement adopté ici, même ce soir. Merci donc Madame Bertrand, de l'avis de la commission. Donc, cet amendement, je trouve que c'est une demande assez générale sinon vague et c'est pour ça que la commission a une nuit. La partie. Merci monsieur le ministre, amis du gouvernement. tout ce qui s'est passé en terme de et de méthode et de contenu sur l'accord Union européenne-Canada a fait en sorte aussi que on s'est fixé de nouveaux objectifs que on veut pas s'arrêter à cette génération de traiter et que on on veut avoir une ambition encore plus élevé et donc on souhaite effectivement inclure dans les, dans les accords à l'avenir ces références systématiques à l'accord de Paris a un certain nombre de, de, de, de règles auxquelles nous sommes attachés effectivement que cela puisse être pris en compte dans les mandats de façon générale, donc nous nous retrouvons assez bien dans l'esprit, en tout cas, en tous les cas qui a présidé à la rédaction de l'amendement, donc avis favorable. Merci donc qu'est ce qu'il y a des explications de vote, s'il n'y a pas d'explication de vote sur cet amendement, je le mets aux voix qui est favorable. Qui compte 3 personnes, donc l'amendement est adopté, c'était le dernier amendement donc je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution européenne sur l'ensemble de cette résolution est-ce qu'il y a des explications de vote.

lorsque sous les débats, on se pose toujours la question de la tradition politique d'une telle résolution, et je crois surtout ce soir, ce qui est important Monsieur c'est d'entendre le message porté par les parlementaires autour de de la situation agricole, nous sommes à la veille de de du l'ouverture du salon Nike demain pour la République, va recevoir 1000 jeunes agriculteurs à l'Élysée, on voit bien aujourd'hui que dans nos territoires, les auditeurs sont remontés ça sur une situation extrêmement compliqué et dans ce contexte nous abordons ce débat qui apporte aussi d'autres situations d'autres difficultés, donc je crois que il faut surtout entendent ce soir le message d'une vraie volonté à la fois d'accompagner ces accords, mais surtout à une volonté de faire en sorte que notre écriture puisse en tirer un bénéfice réel et pas simplement une théorie avec des grands chiffres hé bien une traduction dans les territoires, voilà donc, c'était le message que je souhaitais porter donc au nom de groupe des républicains ne voteront de résolution voilà merci. Monsieur Mulliez, merci, pas d'autres explications de vote. Très brièvement, Monsieur le Président Monsieur Mimi, chers collègues, moi, je voudrais faire 3 remarques : la première, me réjouir de la qualité du débat de la qualité du travail entre la commission des affaires économiques et de la commission des Affaires européennes sur ce point précis d'une milice, nous aurons l'occasion de nous revoir sur ce sujet parce que je souhaite qu'il soit récurrent,

au cours des débats, je pense qu'il il y a aussi danger en ce qui concerne les crédits de la politique agricole commune, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on sous-entend est-ce qu'on sous-entend quelquefois fois plus important que ce que l'on entend

hautement stratégique au moment où tous les États continents qui sont nos concurrents sont en train d'augmenter leur concours publiques à l'agriculture, l'Europe serait en train de diminuer et ça si vous voulez, c'est en quelque sorte une rupture historique, je l'ai dit, pour ceux qui sont assez près des des domaines agricoles la désespérance commence compte les yeux se taisent et on et on commence à voir dans les campagnes, vraiment des gens assez désespérée, le 3ème point dans les accords qui qui qui ont lieu, qui auront lieu peut-être encore demain, il y a une filière qui est fragile qui la filière viande rouge. Globalement, c'est 300000 tonnes que l'Union européenne, mais je dirais rappelons-nous, il y en a quand même 100000 tonnes qui correspondent aux quotas britannique et il faudra se battent pour que les Anglais repartent avec leur 100000 tonnes, vous m'avez compris si vous voulez, il y a d'autres enjeux sur d'autres terrains, mais qui impacteront directement les filières merci. Donc, Monsieur le Président merci donc pas d'autre explications de vote, donc je mets aux voix à l'ensemble de la proposition de résolution européenne qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc cette résolution et t'adopter, je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents, elles sont donc adopté avant de lever la séance, je vous donne l'ordre du jour du jeudi 22 février de 14 heures 30 dans le cadre de l'or du jour réservé au groupe RDSE, une proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité aux fonctionnaires et une proposition de loi sur le régime de l'exécution des peines, des auteurs de violences conjugales, la séance est levée.